La mort de George Floyd, victime de violences policières, a fait se lever un vent planétaire pour dire que les vies noires comptent. Cette exigence trouve un puissant écho en France avec l'affaire Adama Traoré, pour lequel vérité et justice sont exigées. L'impunité doit cesser. Depuis longtemps, les violences policières sont une préoccupation dans les quartiers populaires, mais il a fallu les répressions violentes des gilets jaunes pour que cette préoccupation Les traitements discriminatoires existent au sein de la police, comme au sein de la société, à la nuance près tout de même que les policiers sont détenteurs de l'autorité publique et de la violence légitime, que certains rendent illégitime. Dois-je rappeler toutes ces affaires sordides de violences policières sur fond de racisme ? Certains ont été agressés- Théo hier, Gabriel aujourd'hui -, d'autres ont trouvé la mort- Zyed et Bouna, Adama -, sans compter tous ceux qui sont usés de devoir justifier leur identité, parfois plusieurs fois par jour. Monsieur le Premier ministre, quelle réponse structurelle

je réponds bien volontiers à la question que vous posez parce que, au fond, elle est au coeur du pacte républicain. Comment, dans une société démocratique et libre, peut-on faire prévaloir l'ordre public ?

Ce n'est pas une question simple, madame la présidente. Si nous vivions dans un monde idéal et s'il suffisait de proscrire, d'interdire le racisme, nous l'aurions déjà fait et la loi aurait déjà produit ses effets. Ce n'est pas le cas.

rester calmes en toutes circonstances, appréhender les malfaiteurs, ils sont exposés à un risque permanent du simple fait qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique, bien souvent du simple fait qu'ils portent un uniforme. Nous avons tous en tête exemples de femmes et d'hommes, quels qu'ils soient, qui ont été attaqués et pris pour cible parce qu'ils portaient cet uniforme, qui fait leur fierté et qui est notre protection. Vous avez évoqué cette période particulière et, au fond, malheureuse dite « des gilets jaunes ». Vous avez indiqué, madame la présidente, que cette période démontrerait à l'évidence des violences ...

de violences choisies et exercées par la police sur des manifestants pacifiques. Je vous le dis comme je le pense et comme je l'ai vécu, madame la présidente : nous avons assisté durant cette période-

Je ne veux pas que le débat intense et délicat de la formation, de l'explication des missions de la police, de la définition des techniques les plus adaptées dans une société qui devient de plus en plus violente soit confisqué par des prises de position théâtrales,

Je le dis comme je le pense : nous devons être confiants, respectueux et exigeants vis-à-vis des femmes et des hommes qui font vivre la police nationale et la gendarmerie. C'est cette ligne, qui est une ligne d'équilibre, est une ligne d'équilibre, que je veux tenir, mais je ne veux pas, madame la présidente, que la peur change de camp. Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend,

Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre police et notre gendarmerie républicaines doivent garantir la paix civile et protéger nos libertés, notre égalité et notre fraternité. C'est une immense et noble tâche, accomplie dans des conditions de travail inacceptables, et qui comporte des risques. Nous leur avons unanimement rendu hommage, et pensons

Le reconnaître sans le minimiser, ne jamais couvrir de tels propos ou de tels actes, les punir promptement est une condition de la confiance à restaurer à l'égard d'une grande partie de la jeunesse. C'est un impératif pour la dignité de la police elle-même et pour notre République. Tout commence, monsieur le Premier ministre, par l'arrêt du déni. Un pas dans ce sens a été fait par le ministre de l'intérieur, par vous-même encore tout à l'heure, et nous nous en félicitons. Mais l'ambiguïté subsiste quand on entend M. Nunez parler de nouveau de quelques cas isolés. Nous craignons que, une fois l'émotion passée, on n'en revienne à l'« avant », comme trop souvent dans le passé. Bien entendu, je le répète, pas de faux débat ! En France, la police en tant qu'institution n'est pas raciste,

Que comptez-vous faire pour encourager la remontée de tous les faits répréhensibles, pour vous opposer à la loi du silence et faire passer la loi de la République, pour valoriser dans les formations et dans les carrières celles et ceux qui brillent

l'enseignement supérieur, à l'heure où la crise sanitaire a entraîné la fermeture de nombreuses frontières dans le monde entier, la plupart des étudiants ont dû renoncer à leur séjour à l'étranger. Pourtant, en ce mois de juin, les inscriptions sont en cours de finalisation et l'avenir des échanges internationaux reste incertain pour les étudiants et leurs établissements d'accueil. De nombreuses écoles de formation supérieure prévoient dans les cursus un stage ou une année de césure à l'étranger, mais les étudiants français font face à de nombreuses restrictions en matière de visas, en particulier aux États-Unis, ou bien se voient proposer des stages en visioconférence. Dans le cadre du programme Erasmus, certains étudiants ont dû écourter, ou annuler pour 25 % d'entre eux, leur séjour. À l'inverse se pose la question de l'attractivité de la France à l'égard des étudiants internationaux. Pour certaines grandes écoles, telles que HEC ou Sciences Po, ceux-ci représentent près de 50 % des effectifs. Or la France est passée de la quatrième destination étudiante à la cinquième, derrière l'Allemagne. Le plan Bienvenue en France, qui vise un objectif ambitieux, celui d'accueillir 500 000 étudiants étrangers en 2027, risque malheureusement d'être mis à mal. De nombreux chantiers sont encore à engager. Je pense aux conditions de logement que la période de confinement a mises en évidence. Nous ne pouvons laisser se profiler une année blanche de la mobilité. Les échanges internationaux d'étudiants sont un déterminant important pour notre économie, à la fois gage de dynamisme intellectuel, source d'innovations et de richesse culturelle. Il s'agit donc aujourd'hui de rassurer les candidats internationaux. Madame la ministre, quels dispositifs comptez-vous mettre en place, afin de lever toutes les contraintes actuelles et d'accueillir les étudiants internationaux dans les meilleures conditions ?

vous avez raison, la préoccupation est mondiale et la mobilité, qu'il s'agisse de celle des étudiants ou de celle de l'ensemble des citoyens du monde, est en ce moment empêchée à cause de la pandémie que nous connaissons.

partout dans le monde, dès que possible. J'en veux pour preuve l'organisation des universités européennes à l'intérieur de l'espace Schengen, qui faciliteront le

avons décidé d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir la production de formations à distance, de sorte que les enseignements puissent commencer et être dispensés

de l'Europe et des affaires étrangères, afin d'ouvrir des lieux d'accueil pour les étudiants qui n'ont pas tous les moyens de se connecter là où ils habitent. Ainsi, nous cherchons à préserver l'attractivité de la France et des formations françaises auprès des étudiants internationaux. Le plan Bienvenue en France

Républicains. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, je vous ai entendu parler d'« écroulement ce terme ne m'avait pas choqué. Vous parliez alors d'un écroulement économique et social ; aujourd'hui, la menace qui est devant nous est celle d'un écroulement civique. Comment, en quelques jours, avez-vous pu laisser l'État autant reculer ? des manifestations interdites et, surtout- surtout ! -, vous avez laissé faire des minorités agissantes qui, sous prétexte de l'antiracisme, veulent propager la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre et fracturer notre modèle républicain. Quand une garde des sceaux s'immisce dans une affaire privée, alors qu'elle doit être le garant de l'indépendance de la justice, c'est évidemment l'État de droit qui est fragilisé. Quand, en réponse à son invitation imprudente, elle se voit infliger un camouflet calculé, c'est toute la République qui est humiliée ! Quand votre ministre de l'intérieur

jungle et la possibilité compromise, demain, de la concorde civile. Quand le même ministre fait cette trouvaille, cette acrobatie sémantique de « soupçon avéré », qui va livrer nos policiers et nos gendarmes

les policiers et les gendarmes sont notre bouclier. Vous ne pouvez pas simplement nous dire, tout en leur proclamant votre respect et votre estime, qu'ils sont effectivement pour nous une protection : vous devez le leur prouver ! Reprenez-vous à votre compte

C'est la raison pour laquelle, vous sachant précis, je suis surpris par un certain nombre des expressions que vous avez utilisées dans votre intervention. J'ai du reste essayé de les noter pour ne pas pour ne pas m'exposer à la même critique que celle que je pourrais éventuellement formuler. Vous avez dit, monsieur le président Retailleau, que la garde des sceaux avait voulu s'immiscer dans une affaire privée.

À ce titre, je salue le prêt de 7 milliards d'euros accordé à Air France. Cette aide est significative, mais aussi nécessaire, afin que l'entreprise puisse affronter les difficultés financières du secteur, tout en répondant à des enjeux environnementaux plus que jamais incontournables. Mais Air France ne doit pas oublier que ce secours lui est apporté parce que l'entreprise répond à une obligation de service public en offrant une desserte entre la capitale et les territoires ruraux ou ultramarins. Or, dans ces départements, je constate que la participation à l'aménagement du territoire, attendue, n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas normal, par exemple, que, au mois de juin, les Pyrénées-Atlantiques ne bénéficient que de deux vols quotidiens entre Biarritz et Paris ou, pis encore, pis encore, de deux vols hebdomadaires entre Pau et Paris, voyage qui requiert cinq heures de train. Je regrette que, malgré les sollicitations répétées des parlementaires, Air France n'ait pas augmenté la cadence des vols desservant ces territoires enclavés ou éloignés. Ceux-ci ont pourtant cruellement besoin de liaisons aériennes plus fréquentes dans le cadre de la reprise économique. En effet, comme l'a clairement établi la mission d'information du Sénat sur le rôle du transport aérien dans l'aménagement du territoire, certaines lignes sont vitales pour assurer un désenclavement. Monsieur le secrétaire d'État, je ne peux pas croire que l'État tolère cette situation. Aussi, pouvez-vous me dire comment il compte agir en tant qu'actionnaire d'Air France, et après l'effort consenti pour sauver cette entreprise, afin de la pousser à desservir dignement les territoires qu'elle semble délaisser ? La parole

Durant le confinement, vous le savez, les restrictions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont impliqué une réduction de 95 % des vols. La reprise du trafic intérieur s'organise progressivement depuis le 2 juin, grâce notamment à la levée de la restriction liée à la règle des 100 La majorité des aéroports rouvriront aux vols commerciaux d'ici à l'été. À date, l'offre s'établit à environ 20 % du trafic habituel, avec une augmentation progressive : 35 % en juillet, environ 40 % en août, grâce en particulier à la réouverture de l'aéroport de Paris-Orly, prévue le 26 juin prochain. Nous portons bien évidemment une attention particulière aux lignes d'aménagement du territoire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement. Concernant plus spécifiquement la desserte de Pau, je tiens d'abord à vous rappeler qu'il s'agit d'une ligne commerciale et non pas d'une ligne soumise à obligation de service public plusieurs compagnies opèrent des vols depuis cet aéroport en fonction de la demande : Air France, vous l'avez dit, qui a prévu de programmer deux vols par semaine d'ici à la fin du mois, puis deux cents vols au mois de juillet à destination des aéroports Paris-Orly et de Paris-Roissy ; ASL Airlines, quant à elle, a annoncé la mise en place de quatre liaisons hebdomadaires vers Paris. S'agissant d'Air France, vous savez que la compagnie prépare actuellement un plan de restructuration de son offre commerciale, et le Gouvernement sera vigilant à qu'il ne se fasse pas au détriment des territoires. J'ai d'ailleurs demandé à la direction d'Air France d'entamer très rapidement une concertation approfondie avec les élus concernés.

la crise sanitaire que nous traversons a et aura un impact évident sur les ressources et les dépenses des collectivités territoriales, notamment sur leurs investissements, ce que souligne et regrette déjà le monde économique de nos territoires. C'est pourquoi il est indispensable d'accompagner et de soutenir les investissements de ces collectivités, qui représentent, rappelons-le, 70 % de l'investissement public civil. Le Gouvernement et vous-même, madame la ministre, qui connaissez particulièrement bien les contraintes des petites communes, avez entendu cet appel en lançant des mesures d'urgence en direction des collectivités territoriales. Le troisième projet de loi de finances rectificative de l'année, présenté ce matin, précise ce soutien inédit de l'État vis-à-vis des mécanismes et des garanties. À ce titre, nous saluons le renforcement de l'enveloppe de la dotation de soutien à l'investissement local de 1 milliard d'euros, si utile pour le financement des projets des petites communes. Par ailleurs, une circulaire a été adressée aux préfets, il y a un mois, pour proposer des souplesses dans l'utilisation des crédits d'investissement déjà mobilisés. compte tenu de l'ampleur de la crise économique qui touche les collectivités, ces mesures appellent des précisions sur la façon dont le Gouvernement entend encourager et soutenir les investissements des collectivités. Pour ce qui concerne les projets d'investissements en cours, comment les reliquats de crédits pourront-ils être réalloués à d'autres projets et comment pourront être réaffectées les attributions de subventions ? Plus encore, les collectivités territoriales se demandent quel sera l'engagement du Gouvernement sur la durée. Pourront-elles compter sur ce soutien non seulement pour 2020, mais aussi pour 2021, année qui sera, n'en doutons pas, très difficile également compte tenu de la structure des recettes pour certaines collectivités ? Madame la ministre, je vous remercie de vos réponses, attendues, je le sais, par les élus qui doivent gérer un exécutif local. un exécutif local. La parole est à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, comme vous le rappelez vous-même, les collectivités territoriales portent la majeure partie de l'investissement public et constituent donc un partenaire très important pour les entreprises puisque leur investissement est un levier pour le développement de celles-ci, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, comme nous le savons tous. La réussite de la relance de l'économie, comme vous le dites vous-même, passera donc aussi par les collectivités territoriales. Il est par conséquent très important que ces dernières aient les moyens d'investir. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé il y a dix jours que la dotation de soutien

Ce matin était donc présenté en conseil des ministres le troisième projet de loi de finances rectificative, dans lequel figurent des mesures d'urgence pour les collectivités. La mission qu'a menée notre collègue de l'Assemblée nationale Jean-René Cazeneuve a estimé à environ 7,5 milliards d'euros les pertes de recettes des collectivités, d'euros pour les communes, 3,4 milliards d'euros pour les départements et 0,9 milliard d'euros pour les régions. Vous nous proposez des outils intéressants pour aider les collectivités : clause de sauvegarde- nous l'espérons conforme au principe de péréquation -, soutien aux trésoreries. Mais il me semble qu'on peut s'interroger sur le montant des aides proposées. Pour les communes, les aides financières s'élèvent, si je comprends bien, à 1,75 milliard d'euros, alors que l'estimation des pertes retenue par le Gouvernement est de 3,2 milliards d'euros. L'Association des maires de France considère, pour sa part, que les pertes et les dépenses engagées s'élèveraient à 5 milliards dont 2,2 milliards d'euros de recettes tarifaires, c'est-à-dire les revenus liés à la restauration scolaire, aux transports, aux crèches ou aux piscines. Celles-ci seront-elles compensées par l'État ? Pour ce qui est des départements, une aide plus importante de 2,7 milliards d'euros est annoncée. Permettra-t-elle de compenser intégralement les dépenses sociales engagées pendant la crise ? aucune annonce n'a été faite pour les régions, au grand mécontentement des présidents, qui estimaient, dans une tribune parue dans du 28 mai, à 1,7 milliard d'euros les dépenses exceptionnelles engagées et appelaient l'État à leur donner des garanties, afin de renforcer leurs responsabilités. j'ai bien conscience que plusieurs interrogations figurent dans ma question, mais je peux les résumer de la manière suivante : quels critères avez-vous retenus pour arbitrer la répartition des moyens entre les différents blocs ; pouvez-vous garantir que l'aide de l'État sera suffisante pour qu'aucune collectivité ne soit laissée en difficulté ?

à la moyenne des trois derniers exercices, l'État versera une dotation permettant de garantir ce niveau. Aucun critère, aucune démarche ne limitera l'activation de ce filet de solidarité. Autrement

des régions, le calendrier est un peu différent, car la loi prévoit déjà des mécanismes de garantie sur les recettes 2020, qui conduiront l'État à leur compenser environ 500 millions d'euros, en particulier la baisse des rentrées de TVA.

soit une semaine après la publication par d'une étude sur l'usage de l'hydroxychloroquine, votre ministère a interdit le recours à celle-ci dans le traitement du Covid-19. Cette interdiction faisait suite au décret du 25 mars, qui défendait aux médecins libéraux de prescrire cette molécule à leurs patients. On sait ce qu'il est advenu de cette étude, qui a été désavouée d'abord par les éditeurs du, et ensuite par trois de ses quatre auteurs. Elle était en réalité une vaste farce dont les scientifiques, les soignants, les patients et votre gouvernement ont été les dindons C'est triste ... On me rétorquera que d'autres études n'ont pas pu démontrer l'efficacité de cette molécule, mais la vérité est que les protocoles mis en concurrence sont tellement divergents qu'il est impossible d'affirmer aujourd'hui que cette molécule est efficace ou pas, même s'il semble que les patients traités dès leur dépistage et dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation s'en sortent majoritairement mieux. Une chose est absolument certaine, en revanche seuls les médecins sont aptes à prescrire le protocole qui leur semble le mieux convenir à leurs patients. Votre gouvernement a peut-être un goût certain pour les ordonnances ; moi, je préfère celles qui portent un caducée ! Ma question est simple, madame la secrétaire d'État ne serait-il pas temps de reconnaître qu'il y a eu de l'emballement dans cette affaire et de redonner aux médecins la liberté de prescrire ? Très

De nombreux travaux de recherche- vous en avez cité quelques-uns -ont été menés pour tenter d'analyser son efficacité et son innocuité dans le traitement du Covid-19. Le ministre et l'ensemble du Gouvernement ont été transparents : tous les efforts ont été accomplis, afin de trouver des réponses rigoureuses et scientifiques à cette question. À ce jour, les travaux de recherche conduits n'ont pas réussi à démontrer avec un niveau de preuve suffisant l'efficacité de l'hydroxychloroquine chez les malades hospitalisés ou dans les formes les plus simples Par ailleurs, de nombreuses études ont montré des effets secondaires connus et renforcés dans le cas de certaines associations médicamenteuses. Les résultats de deux travaux scientifiques- issus d'auteurs similaires -ont dû être retirés en raison de questions sur leur intégrité scientifique. Nous le déplorons. Néanmoins, l'ensemble des études rassemblées à ce jour sur la question

dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin

l'entreprise Luxfer produisait des bouteilles d'oxygène ; l'entreprise Famar, de la chloroquine ; Péters Surgical, des sondes de Montin pour les intubations la sucrerie de Toury, en Eure-et-Loir, du sucre et de l'alcool nécessaires aux gels hydroalcooliques. Mais il y a aussi l'entreprise Peugeot Japy, à Valentigney, qui a été brutalement fermée hier Il y a aussi General Electric, qui vient de connaître 40 000 heures de travail délocalisées en Chine ! Des dizaines et des dizaines d'entreprises sont au bord du dépôt de bilan,

sixième puissance économique mondiale, était incapable de produire sur son territoire des masques, des combinaisons de protection, des tests biologiques, du gel hydroalcoolique, des respirateurs, des médicaments. Jérôme Fourquet disait

aujourd'hui à la France comme endroit pour investir, puisque notre pays est toujours la première destination pour les projets industriels soutenus par des partenaires étrangers, selon les résultats que vient de publier le cabinet Ernst&Young.

menons une politique industrielle au service de la santé. Nous aurons de beaux projets à vous présenter dans les prochains jours. la Chine ne peut pas être l'usine du monde ! Il faut que nous ayons la volonté de produire dans notre pays. À force de tout expliquer, à force d'avoir accepté les délocalisations, on s'est aperçu, durant cette crise très difficile, que la France pouvait devenir une nation de seconde zone. Il n'y a rien de pire ! Il est temps de réagir. Veillons, avec les collectivités locales, avec le Comité chaque fois qu'une entreprise est en difficulté, elle reste sur notre territoire. Nous avons besoin d'emplois industriels, nous avons besoin d'emplois tout court, nous avons besoin d'une France industrielle, une France de producteurs, pas seulement de consommateurs. de consommateurs. Je salue Martial Bourquin, qui va quitter le Sénat pour rejoindre sa commune d'Audincourt, qui a bien de la chance de le retrouver. Je veux saluer son engagement pour le Sénat, notamment sa persévérance sur les questions industrielles et d'emploi. La parole est à Mme Claudine Thomas, pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame la ministre, cette année, 658 000 lycéens attendaient le verdict de Parcoursup. Dès les premiers résultats connus, les plaintes se sont multipliées, rappelant les nombreux ratés qu'avait déjà connus ce dispositif l'année dernière. Les améliorations promises par votre ministère ne sont manifestement pas au rendez-vous. Pour tenter d'accepter ce qui apparaît comme arbitraire, il faudrait au moins avoir des éléments pour comprendre les critères de sélection. Mais rien n'est plus opaque que la façon dont l'interface prend ses décisions.

Parcoursup avait pourtant été mis en place pour permettre un système plus juste. Or, dans certaines universités, la sélection passe encore par une forme de tirage au sort sans doute plus technologique, mais tout aussi injuste. Ces dernières, incapables de traiter correctement et individuellement les dossiers, ont mis en place des algorithmes pour classer et évaluer les candidats. En plus de pénaliser des lycéens méritants, cela conduit à standardiser le profil des candidats. Les conclusions de la Cour des comptes, dans son rapport de février dernier, vont dans le même sens. La Cour a en effet souligné le manque de transparence, l'aspect uniforme des dossiers, l'automatisation croissante du système. Elle note également que la motivation des élèves n'est pas prise en compte et conclut que les performances de Parcoursup ne sont pas meilleures que celles de l'antique système ! Le Gouvernement avait affiché sa volonté de remettre de l'humain dans le système de l'orientation et de l'inscription à l'université. La réalité est malheureusement tout autre. Madame la ministre, qu'envisagez-vous de faire pour remédier à cette situation d'injustice criante ?

pour accompagner et orienter les lycéens- cela ne se faisait pas à l'époque d'APB -, au regard du travail qui est conduit dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur pour étudier les dossiers et faire des propositions-

par les professeurs, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. Madame la sénatrice, cette année, 2 % de voeux supplémentaires ont été exprimés par les lycéens, malgré la période de confinement,

plus tôt que les années précédentes, pour que, là encore, nous puissions mieux accompagner les candidats avant même l'obtention de leur baccalauréat. Alors oui, madame la sénatrice, je l'ai toujours dit : ce dispositif a vocation

parfois des difficultés, et bien sûr nous travaillons à les résoudre chaque jour. J'en veux pour preuve le fait que nous comptons 20 % de boursiers supplémentaires ; j'en veux pour preuve que

Du point de vue financier, cette annonce répond aux très fortes inquiétudes d'un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire et par ses conséquences économiques. Je salue la réactivité du Gouvernement sur ce sujet capital. Cette enveloppe est volumineuse, c'est vrai, mais elle doit surtout être efficace pour préserver l'emploi dans nos territoires. Vendredi dernier, l'entreprise Daher, spécialisée dans l'équipement aéronautique, annonçait un plan de restructuration concernant ses deux sites de Montrichard et Saint-Julien-de-Chédon, dans mon département, le Loir-et-Cher. Avec une baisse de 40 % de son chiffre d'affaires

soutenir et relancer la filière aéronautique, il faut commencer par sécuriser les investissements industriels du secteur et l'emploi local, et ce pour toutes les entreprises du secteur aéronautique, des équipementiers jusqu'aux compagnies aériennes. Il est essentiel de donner à des entreprises comme Daher de la visibilité et des éléments concrets de soutien pour les aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix stratégiques et à ne pas s'engager dans une restructuration trop lourde sur le plan de l'emploi. peut-il nous détailler les modalités de ce plan de relance et nous garantir que la priorité sera la préservation de l'emploi, pour Daher comme pour les autres entreprises du secteur aéronautique ? La

et qui permettent à la France d'être le seul pays, avec les États-Unis, à pouvoir construire un avion de A à Z. Cette filière est un fleuron de notre industrie et nous devons

que l'aviation commerciale est clouée au sol. Il s'agit d'accompagner cette industrie pour que, demain, face à la concurrence américaine et chinoise, elle soit au rendez-vous et puisse rebondir.

dans le cadre de la reprise progressive des cours à l'école, votre dispositif sport-santé-culture-civisme, dit 2S2C, entend offrir des activités éducatives sur le temps scolaire. Il est conçu comme une réponse à la crise sanitaire et aux contraintes du protocole, qui entraînent des conséquences très lourdes quant au nombre d'élèves pris en charge. Nous le savons tous : l'absence de reprise scolaire pour une part non négligeable des élèves est constatée et regrettée de manière unanime. Les dangers de la déscolarisation physique sont immenses et les dégâts seraient irréversibles si la majorité des enfants ne retrouvaient pas le chemin de l'école avant le mois de septembre prochain. Hier encore, le maire de Besançon me demandait d'intercéder auprès de vous pour un desserrement du protocole sanitaire ; alors que les parcs sont désormais ouverts, les écoles, aujourd'hui, ne le sont pas totalement.

! Je sais que ce dispositif, insuffisamment financé, sera, surtout en zone rurale et parfois en zone urbaine, source d'inégalités. La sollicitation des finances locales ne saurait devenir le moyen ordinaire de mise en oeuvre budgétaire de votre gouvernement.

: il a fallu le courage du Président de la République pour le décider le 11 mai dernier. Aujourd'hui, tout le monde constate que c'était la bonne décision. D'une certaine manière, c'est un hommage que vous nous rendez en nous demandant d'accélérer !

ma collègue Josiane Costes vous a déjà fait part de ses craintes, et ces dernières semblent se confirmer. En effet, dans un communiqué récent, Air France et sa filiale Hop ! ont annoncé vouloir réduire de près de 40 % leurs vols régionaux d'ici à 2021. Une telle décision frappe une nouvelle fois de plein fouet des territoires déjà durement éprouvés. Vous l'avez compris : nous ne pouvons accepter des décisions unilatérales pénalisant de nombreux bassins économiques et industriels.

Quelles contreparties allez-vous exiger de cet opérateur monopolistique ? Les OSP seront-elles bien identifiées comme un enjeu stratégique essentiel au développement des territoires ? Comment comptez-vous mesurer les niveaux de soutenabilité acceptables pour rouvrir ces lignes ? Enfin, laisserez-vous les collectivités seules négocier avec Air France, toujours plus prompt à alimenter les procès en non-rentabilité de ces lignes, au mépris du service qu'elles rendent aux territoires, et sans afficher clairement les exigences de l'État ? L'État reste le garant de l'aménagement et de l'égalité des territoires. Pour les Hautes-Pyrénées, le Cantal ou la Lozère, l'avion demeure le seul salut. Nous le savons tous pertinemment, nos territoires enclavés et éloignés ne bénéficieront jamais de lignes de

La relance du pays ne se fera qu'avec un soutien ambitieux des collectivités. Face à la crise, les élus locaux ont assumé un rôle essentiel pour pallier les manques et assurer la continuité de l'État. On ne pourra pas se contenter de soutenir la

Certaines estimations dépassent même les 10 milliards d'euros. Les départements, en première ligne pour la solidarité, accumulent les pertes, mais ils ne bénéficieraient que d'une avance sur les droits de mutation : l'effet de ciseaux budgétaire promet d'être redoutable.

Madame la ministre, ce plan de soutien n'est qu'une compensation, alors que les collectivités territoriales peuvent être un vecteur puissant de la relance : quels véritables moyens allez-vous mettre à leur disposition ?

en particulier dans le domaine militaire, l'un des marqueurs de son quinquennat, ainsi que la boussole de son action européenne. Le déploiement d'un fonds européen de défense ambitieux devrait en être la concrétisation et le symbole. Comment devons-nous interpréter ce revirement ? Quelles en sont les conséquences pratiques et opérationnelles, notamment pour l'industrie de la défense, dans le cadre du plan de relance ?

d'euros : c'est un progrès, mais, je vous l'accorde, le compte n'y est pas encore. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous avons écrit au Haut Représentant de l'Union européenne, ainsi qu'à nos homologues européens, afin que le fonds européen de défense puisse être porté à un niveau ambitieux. Ce dispositif est plus que jamais nécessaire. La crise du Covid a montré que nous avons besoin de plus d'Europe, de plus de souveraineté européenne. Le fonds européen de défense devra donc également prendre sa part de la relance économique, dont nous avons besoin collectivement au sein de l'espace européen.

nous voulions. Nous n'avons pas réussi à convaincre ; nous étions seuls ; nous pensions être les meilleurs ; et aujourd'hui nos partenaires européens ont du mal à entendre la voix de la France et à nous suivre. Je compte sur vous pour améliorer les choses ! Mes

Mes chers collègues, la commission des lois demande que le délai limite de dépôt des amendements de séance sur le projet de loi organique portant report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles soit reporté du lundi 15 juin au mercredi 17 juin à douze heures. La commission se réunira à l'issue de la discussion générale pour l'examen des amendements de séance. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place en mars dernier. J'invite chacune et chacun d'entre vous à veiller au respect des distances de sécurité.

En ces termes délicats qui sont propres à l'administration fiscale, Bercy- appelons les choses par leur nom -voulait pouvoir prescrire qu'un certain nombre d'organismes déposent leur trésorerie au Trésor public,

l'article était tellement large qu'il était impossible de savoir quels organismes seraient sollicités. En particulier, des organismes privés chargés d'une mission de service public pouvaient se trouver dans cette situation,

Un tel accord n'aurait sans doute pas été possible sans la disponibilité, l'écoute attentive et la démarche d'emblée constructive de Mme la rapporteure de la commission des lois. Je sais, madame Jourda, que le sentiment que j'exprime à cet instant est partagé par votre homologue à l'Assemblée nationale. Permettez-moi de remercier également M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, dont l'expertise et la rigueur ont permis au Gouvernement d'affiner les dispositifs qu'il envisageait. Nous avons avancé ensemble vers des solutions, parfois introduites en urgence, pour notre économie et pour la préservation des emplois et des compétences.

mais au sein même des groupes politiques. Dans ces conditions, il semblait important d'entendre les doutes que ces clivages exprimaient. Ce souci du dialogue auquel j'ai tenu et auquel je sais votre assemblée particulièrement attachée a porté ses fruits : les accords trouvés sont satisfaisants pour tout le monde. Ainsi, l'article 3, relatif à la centralisation de certaines trésoreries, précise un peu plus encore quels organismes sont exclus du dispositif, à commencer par les caisses de retraite, les Carpa et un certain nombre d'établissements sociaux et médico-sociaux. Au terme de ce parcours

Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, « la France gouvernée par une assemblée unique, c'est l'océan gouverné par l'ouragan », écrivait Victor Hugo. ! Véritable gage de démocratie, le bicamérisme garantit l'existence d'une authentique discussion législative, qui privilégie l'esprit de sagesse et concourt à la qualité de la loi. Le présent texte en est la parfaite illustration la rédaction adoptée en commission mixte paritaire est assez éloignée de celle présentée en conseil des ministres, notamment par le nombre de ses articles et celui des habilitations à légiférer par ordonnance. Particulièrement attaché au débat parlementaire, comme nous tous, je me félicite que nos deux assemblées se soient entendues pour permettre au Parlement de conserver ses prérogatives de législateur en limitant fortement les habilitations aux seuls cas où elles sont indispensables. Nous sommes ainsi passés de quarante habilitations à dix ... La crise sanitaire que notre pays traverse est d'une ampleur inédite, et son impact sur notre économie sera considérable. Selon les dernières prévisions de la Banque mondiale, publiées avant-hier, le PIB mondial devrait se contracter de 5,2 % en 2020 ; et c'est dans la zone euro que le recul sera le plus marqué. Hier, la Banque de France a annoncé une récession d'environ 10 % cette année et estimé que le taux de chômage atteindrait plus de 10 % à la fin de 2020, pour s'envoler à 11,5 l'année prochaine. Les effets de la pandémie devraient se faire sentir pendant deux ans. Aussi, mettre en place les moyens d'affronter cette crise sans précédent et d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens relève d'une impérieuse nécessité. Pour répondre à ces enjeux, sénateurs et députés de la commission mixte paritaire ont travaillé en bonne intelligence, dans l'intérêt des Français, ce qui a permis d'aboutir à un compromis. Les sujets de désaccord étaient nombreux, mais l'échec annoncé de la commission mixte paritaire n'a finalement pas eu lieu, ce dont nous nous félicitons. Pourtant, les conditions dans lesquelles nous avons eu à examiner ce texte en première lecture étaient pour le moins compliquées, comme l'avait souligné notre collègue Josiane Costes : des délais particulièrement contraints

Dans ce contexte, plusieurs dispositions vont dans le bon sens. Je pense notamment au nouveau dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, qui permettra d'accompagner les entreprises durablement affectées par la situation sanitaire et économique. Les entreprises confrontées à une activité encore réduite pourront ainsi, en accord avec les syndicats, diminuer le temps de travail ou les salaires, à condition de maintenir totalement l'emploi. Une aide de l'État compensera une partie de la perte de pouvoir d'achat. Nous saluons également la prolongation des titres de séjour, le maintien des garanties de protection sociale complémentaire, l'ouverture des droits à la retraite des salariés placés en activité partielle et la dérogation aux règles de cumul emploi-retraite pour les soignants, ainsi que l'intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés. nous nous félicitons que la commission mixte paritaire ait retenu certains apports de la Haute Assemblée, comme la meilleure gestion des fonds de commerce pour les entreprises en difficulté, l'allongement d'expérimentations pour favoriser l'insertion des agents handicapés dans la fonction publique et le report de la caducité des règlements locaux de publicité.

de la commission des finances- même si la durée et le champ de l'habilitation ont été réduits. Surtout, nous déplorons l'extension de l'expérimentation des cours criminelles. De neuf départements, le Gouvernement nous proposait de passer à trente ! En première lecture, nous avons rejeté cette extension,

monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite à mon tour de l'accord que nous avons pu trouver le 2 juin dernier, grâce à des concessions réciproques de nos deux assemblées. Sur la forme, l'état d'esprit constructif qui a présidé à l'examen de ce texte est, au risque de me répéter, à saluer. Une démarche collective de clarification a été suivie afin de préserver les droits du Parlement. De cette façon, la grande majorité des dispositions ont pu être directement inscrites dans le projet de loi.

Sur le fond, qu'on le qualifie de « fourre-tout », de « foisonnant » ou de « dense », ce projet de loi a le mérite de répondre à des besoins divers, que cette crise sanitaire inédite a fait naître dans des domaines aussi variés variés que l'économie, le social, l'administration, la justice, la santé. Il comporte des dispositions conciliant protection de l'emploi et accompagnement de la reprise économique et d'autres permettant de garantir la continuité du service public. Je songe notamment au dispositif spécifique d'activité partielle mis en place par accord collectif, au développement de l'intéressement dans les très petites entreprises et à la constitution de droits à retraite du 1 mars au 31 décembre 2020 au titre du chômage partiel, sans oublier l'indemnisation des chômeurs en fin de droits à partir du 1 mars 2020. Je m'attarderai un instant sur les mesures qui concernent les outre-mer et qui, même si elles n'ont pas de lien direct avec la pandémie, n'auraient pas trouvé à s'inscrire dans le calendrier parlementaire à venir, alors même qu'elles sont vivement attendues par nos compatriotes. Je pense à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française, à la prorogation de l'agence des cinquante pas géométriques aux Antilles et à celle de la commission d'urgence foncière à Mayotte.

Repousser encore cette installation, qui a déjà fait l'objet de trois reports, n'aurait pas été acceptable ! Ensuite, je me félicite de la prolongation, à titre exceptionnel et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, de l'indemnisation des demandeurs d'emploi résidant à Mayotte dont les droits sont arrivés à échéance depuis le 1 mars dernier. Cette mesure tient légitimement compte du fait que la période de confinement a été plus longue dans ce département.

a permis de réintroduire l'habilitation relative à la centralisation des trésoreries, dans une rédaction bienvenue qui exclut de son champ d'application plusieurs organismes, tels que les organismes établis par les collectivités territoriales et les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

aux seules procédures contraventionnelles sans victime la faculté donnée aux procureurs de la République de classer sans suite. Je salue également la limitation mesurée de l'extension de l'expérimentation des cours criminelles à dix-huit départements. Mes chers

mes chers collègues, dans sa version initiale, ce projet de loi prévoyait quarante ordonnances, démontrant la volonté du Gouvernement de brider la capacité d'amendement du Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat sont cependant parvenus à modifier les moyens d'action prévus dans ce texte, réduisant de manière drastique le recours à l'article 38 de la Constitution. Malheureusement, force est de constater que, si le Parlement a pu modifier positivement la forme de ce projet de loi, il n'a pas jugé utile d'en améliorer le fond. Face à l'urgence sanitaire, l'exécutif aurait pu se tourner vers une gouvernance apaisée, privilégiant des mesures susceptibles de faire consensus. Nous observons- hélas ! -que le Gouvernement a préféré se servir de la crise économique pour faire avancer son agenda libéral ; en attestent notamment les nouvelles dispositions rendant flexible le recours aux aux contrats à durée déterminée. Ni la récession ni le chômage de masse n'amèneront le Gouvernement à se départir de sa libérale. En ces temps incertains, salariés, employés et ouvriers de France auraient grandement eu besoin de la stabilité d'un Nous notons que vous ne comptez leur offrir que la fragilité d'un contrat à durée déterminée (CDD) renouvelable, alors que de nombreux Français ont pris des risques en première ligne pendant la pandémie. Dans ce texte aux mesures diverses, tout n'est cependant pas à mettre de côté. Des éléments positifs subsistent, concernant notamment la question de l'activité partielle. Nous saluons évidemment la prolongation des dispositifs prévus en la matière dans certains secteurs, en particulier le tourisme et la restauration. le texte validé par la commission mixte paritaire se limite à une demi-mesure qui finira par se heurter à la réalité. Le confinement et l'arrêt de l'économie ont vidé les carnets de commandes de nombreuses entreprises françaises, notamment les PME et les TPE. Beaucoup n'appartiennent pas aux secteurs concernés par la prolongation des dispositifs de chômage partiel, et leurs salariés ne pourront de ce fait en bénéficier. De la même manière, si nous pouvons nous réjouir du choix qui a été fait de prolonger la validité des titres de séjour des étrangers présents sur notre territoire, nous déplorons que les dispositifs mis en place afin d'allonger la durée de travail des étudiants et des travailleurs saisonniers étrangers aient été conditionnés à la durée de l'état d'urgence sanitaire, preuve s'il en est du manque de considération de l'exécutif pour les personnes migrantes. Il est regrettable que, aux yeux du Gouvernement, l'étranger ne bénéficie pas de véritables droits qui ne seraient pas soumis aux besoins d'une conjoncture donnée.

des dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, il n'en a rien été dans les faits, étant donné que vous avez plutôt légiféré sur l'ouverture de la saison de la chasse ou sur l'organisation des fédérations sportives. Nous déplorons donc l'absence criante dans ce texte de mesures sanitaires et sociales, ainsi que de dispositifs ayant trait à la gratuité des masques ou à l'allongement du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse pour celles qui n'ont pas pu y accéder pendant la crise sanitaire. Le texte qui sera voté aujourd'hui fait la part belle à la flexibilisation du droit du travail, tout en mettant à mal le dialogue social. Il précarise les salariés tout en déconsidérant les étrangers. Il va sans dire qu'une telle philosophie n'est pas de nature à nous satisfaire. Pour ces raisons, le groupe CRCE votera contre ce texte. La parole

Tout comme le reste de l'Europe, nous entrons dans une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Les mois qui arrivent seront décisifs, et nous devons donc préparer l'avenir avec des mesures de souplesse. Le texte final a largement repris les dispositions proposées par le Sénat. En réduisant le nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance de quarante à dix, le Parlement s'inscrit dans une logique claire il conserve la prérogative législative et s'assure que toute sa place sera laissée au débat parlementaire. Le Gouvernement sera toutefois habilité à légiférer par ordonnance sur des sujets fondamentaux.

prochain, pourra si nécessaire être allongée. Ainsi, la question pourrait être de nouveau traitée prochainement. La crise que nous traversons a fragilisé notre économie, qui redémarre lentement depuis le 11 mai, mais surtout depuis l'entrée dans cette deuxième phase de déconfinement. Il est donc important de soutenir les entreprises et leurs employés. Qu'elles soient petites ou moyennes, les entreprises sont le coeur de notre tissu économique. À ce titre, les décisions prises concernant l'activité partielle vont véritablement dans le bon sens. Le groupe Les Indépendants a d'ailleurs soutenu des points relatifs au régime d'intéressement, qu'il considère comme un élément central rapprochant les intérêts communs des salariés et des entreprises.

concernant les mesures relatives à l'allocation chômage des intermittents du spectacle, des travailleurs indépendants et des travailleurs à la mission. Il est en effet très important de bien prendre en compte toutes ces situations spécifiques. Je terminerai en soulevant deux points. Le premier concerne la justice de notre pays et son exercice. La commission mixte paritaire a rétabli l'élargissement de l'expérimentation des cours criminelles chargées de juger des crimes sans jury populaire,

Nous sommes donc loin de l'image qui est souvent véhiculée dans l'opinion publique et des critiques parfois exprimées par le pouvoir exécutif- jamais par vous, monsieur le ministre-d'un Parlement trop lent ou d'un bicamérisme redondant, voire inutile. Chacune des deux chambres apporte son expertise et améliore les textes déposés par le Gouvernement. Sans être aux ordres, le Parlement est conscient de sa responsabilité dans la crise traversée. Nous mesurons les enjeux et les contraintes. Sans être aveuglément suiveurs, nous sommes constructifs et nous apportons l'expérience vécue sur le terrain, indispensable à la bonne écriture de la loi et à son adaptation dans une situation qui demande à la fois agilité et réactivité. Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Assemblée nationale et le Sénat ont partagé les mêmes objectifs : limiter le plus possible le nombre d'ordonnances, et donc écrire en clair un maximum de dispositions ; mieux encadrer le champ des habilitations restantes ; limiter au maximum les mesures du texte à des dispositifs dérogatoires répondant précisément à l'état d'urgence sanitaire. Dans ce cadre, le groupe Union Centriste a largement apporté son soutien aux propositions de la rapporteure de la commission des lois, Muriel Jourda, et à nos deux collègues rapporteurs pour avis des commissions des affaires sociales et des finances. Les différentes sénatrices et sénateurs de mon groupe ont apporté leur pierre à la construction législative.

de six mois de la caducité des règlements locaux de publicité de première génération au-delà du 14 juillet 2020, soit une fin de validité le 13 janvier 2021. S'il peut paraître technique, 2021. S'il peut paraître technique, ce report est très utile pour les élus municipaux et intercommunaux qui ont cumulé confinement et report des élections. Il sécurise juridiquement leurs décisions et permet aussi à ceux qui viennent d'être élus ou qui vont l'être de prendre leurs marques.

Par ailleurs, je souhaite mentionner l'adoption d'un amendement de Valérie Létard et des collègues de mon groupe à l'article 1 visant à préciser l'une des rares habilitations restant dans le texte afin de tenir compte de la situation particulière des entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, fermées depuis le 15 mars ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ce secteur, notamment l'amont grossiste. En outre, je dois me faire cet après-midi le relais de nos collègues de la Polynésie française pour deux raisons bien particulières et très liées à leur territoire. Tout d'abord, l'article 1 E relatif au statut des agents contractuels en Polynésie française, supprimé en commission sur l'initiative de Lana Tetuanui, a été rétabli dans une rédaction de compromis reportant uniquement de six mois la réforme du statut de ces agents contractuels.

un amendement ayant pour objet de neutraliser les effets de l'état d'urgence sur la transformation de CDD en CDI dans les trois versants de la fonction publique. En conclusion, madame la présidente, monsieur le ministre, les sénateurs et sénatrices du groupe Union Centriste voteront en faveur du texte établi par la commission mixte paritaire sur ce projet de loi. La parole

le Gouvernement nous conduit à une situation où le Parlement ne fait plus vraiment la loi. Au total, près de soixante ordonnances ont été prises depuis le début de la crise du Covid-19, et c'est extrêmement préoccupant. Le présent projet de loi comptait à l'origine pas moins de quarante demandes d'habilitation à légiférer.

Le Gouvernement a pris l'habitude de tordre les institutions et leur pratique pour les adapter à ses projets et à ses priorités. Il ne se soucie pas que ces dernières ne soient pas partagées par les représentants du peuple, qu'il place dans l'impossibilité matérielle d'accomplir leur mission. C'est une triste performance, qui relève de la même stratégie délétère que celle qui épuise notre hôpital, notre école ou nos services publics ; elle consiste à mettre les institutions qui doivent servir le peuple dans l'impossibilité de faire correctement leur travail. C'est sans surprise que nous sommes obligés de constater que la philosophie de ce texte n'a pas évolué entre la première lecture au Sénat et la rédaction résultant des travaux de la commission mixte paritaire. Les thématiques hétérogènes qu'il traite sont impuissantes à masquer un projet profond- toujours très « ancien monde » -et une méthode imparfaite qui mettent à mal nos fondamentaux. Si mes collègues siégeant sur les travées de gauche et moi-même avons salué des décisions que nous savons coûteuses pour le budget de l'État, mais nécessaires- telles que les mesures de chômage partiel -, nous ne pouvons nous en satisfaire tant ce que propose le présent texte est par ailleurs problématique. il prévoit à la fois des mesures positives et de profondes attaques contre ce qui fait notre État social, singulièrement les acquis des travailleurs. Visant à préserver l'emploi et les compétences dans les secteurs touchés durablement par une baisse d'activité en ajustant notamment la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, la démarche pèche parce qu'elle accroît la pression sur les salariés en jouant sur leur précarisation. Ce texte a notamment pour objet de permettre aux entreprises de modifier le régime des CDD et des contrats de mission. Les dérogations pourraient ainsi être négociées au niveau des entreprises pour tous les contrats courts signés avant la fin de l'année, dans un contexte où la démocratie sociale est déjà très fragilisée. fragilisée. Il s'agit de graver dans la loi une libéralisation du régime des CDD. En matière de justice, nous nous sommes fortement émus de l'absence d'évaluation et de recul sur l'extension de l'expérimentation des cours criminelles. Les modalités de la mobilisation des jurys populaires- par ailleurs intéressante -, nous inquiètent, notamment la possibilité d'une limitation du public pour leur tirage au sort. L'absence de débat parlementaire sur une réforme de la justice des mineurs, reportée par la force des choses, signale aussi une démarche politique à l'emporte-pièce, alors même que des représentants de la magistrature, du barreau ou de la protection judiciaire de la jeunesse appellent à l'abandon de cette réforme extrêmement mal engagée.

considérés dans une logique utilitariste, pour répondre à la demande de main-d'oeuvre agricole, sont autorisés à travailler jusqu'à 80 % du temps, quel qu'en soit l'impact sur leurs études. La manière dont on envisage le rôle de ces jeunes est tout un symbole.

Nous avons choisi de répondre par nos amendements aux besoins d'une population qui voit fondre sur elle les conséquences sociales dramatiques de la crise. Nous avons pris le parti de réintroduire dans ce projet de loi cette dimension sociale qui peine à transparaître dans les textes du Gouvernement. Nos propositions ont porté sur la gratuité des masques et la sécurisation des parcours d'insertion, la prolongation du chômage partiel, la protection des jeunes vulnérables, la sécurisation du droit au séjour, la confirmation du droit à l'interruption volontaire de grossesse, le soutien aux collectivités locales, ou encore le maintien du versement des pensions alimentaires par les caisses d'allocations Alors que le texte accède à l'une de nos demandes- la prise en compte du chômage partiel pour le calcul des retraites -, nous avons voulu que cette mesure permette une véritable préservation du droit à la retraite, y compris pour les carrières courtes, tant pour le nombre de trimestres que pour le montant des pensions.

Le projet que le présent texte dessine en creux témoigne de la difficulté à répondre à l'acuité de la crise sociale qui se profile en fonction des contraintes du réel. Il est particulièrement préoccupant d'observer qu'au sein du Parlement les majorités demeurent arc-boutées sur des modèles passés et dépassés, alors que les situations individuelles des personnes vulnérables ou fragilisées par la crise se dégradent très vite. Dans ce contexte, nous avons besoin d'un fonctionnement institutionnel serein et efficace ; or nous n'en prenons pas le chemin. La propension à produire des textes fourre-tout dans des délais trop courts qui ne respectent pas le travail du Parlement ne répond pas aux attentes démocratiques de nos concitoyens. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste et républicain et les

nous achevons aujourd'hui l'examen d'un projet de loi portant sur des sujets très variés, tournant pour la plupart autour des questions relatives à la sortie de crise sanitaire et de ses implications- pour la plupart car de nombreux sujets sans rapport, comme les conséquences des essais nucléaires ou le Brexit, sont aussi évoqués dans ce projet de loi qui est passé de quarante articles à plus de soixante aujourd'hui. Pour commencer, je tiens à exprimer à mon tour ma satisfaction qu'un grand nombre des dispositions initialement énumérées parmi les ordonnances de l'article

Sur le fond, sans pouvoir couvrir l'ensemble des problématiques traitées par ce texte, je me bornerai à quelques remarques sur certaines des questions qui avaient plus particulièrement retenu l'attention de notre assemblée. Je ne reviendrai pas sur les mesures sociales au sujet desquelles s'exprimera dans un instant mon collègue rapporteur pour avis René-Paul Savary. Premièrement, en plus de la réduction du nombre de d'ordonnances que j'ai déjà évoquée, je souhaite souligner la réduction de la durée des habilitations. Il était impératif de les assortir de délais adaptés et, autant que possible, brefs.

L'article 3, qui prévoit une habilitation portant sur le dépôt des disponibilités de trésorerie de certains organismes, avait été supprimé par le Sénat. Le rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, avait en effet souligné que le domaine concerné était trop large et flou. avec satisfaction que la commission mixte paritaire a trouvé un compromis permettant de mieux délimiter les situations concernées, rassurant ainsi les acteurs et rendant cette habilitation plus acceptable. Je salue également le compromis trouvé sur la question du report de l'entrée en vigueur au niveau territorial du répertoire des représentants d'intérêts. Dans le contexte actuel, mettre en oeuvre ce dispositif à la date prévue serait source de difficultés techniques considérables pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, cela indépendamment de l'intérêt que l'on reconnaît à cette mesure. Permettez-moi également de mentionner la présence dans le texte final de la rédaction issue d'un amendement que j'ai défendu avec mon collègue Loïc Hervé. Ce dispositif facilitera le dépistage du coronavirus par la médecine du travail et prolongera deux

Cependant, durant les travaux de la commission mixte paritaire, il a été possible de négocier une réduction de son envergure. Elle concernera donc dix-huit juridictions au lieu de trente. C'est un pas dans la bonne direction, même s'il ne nous satisfait pas. Par ailleurs, comme le président Philippe Bas l'a souligné, accepter ce compromis dans le cadre des travaux de la commission mixte paritaire ne signifie pas nécessairement approuver cette politique. Pour finir, je tiens à remercier une nouvelle fois les rapporteurs du travail considérable réalisé, qui les a conduits à jongler entre les thèmes très variés. Le texte de cette commission mixte paritaire nous semble acceptable, car il sauvegarde une part substantielle des avancées réalisées par le Sénat. Cependant, nous condamnons une fois de plus la méthode consistant à discuter pêle-mêle

je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Personne ne demande la parole ?

l'Union européenne. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d'un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires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

les électeurs de 30 143 communes de France ont élu des conseils municipaux complets à l'issue du premier tour de scrutin. après un délai dû à la crise sanitaire que nous avons traversée et traversons encore, les conseils municipaux ont pu se réunir, les maires et les adjoints ont pu être élus, la vie locale peut reprendre son cours. Vous aviez

les conséquences : dans ces communes, les exécutifs élus en 2014 sont toujours en place. Dans ces communes, l'économie locale et les grands projets sont en partie suspendus. Dans ces communes, les intercommunalités, si importantes pour la vie de nos collectivités et de nos concitoyens, n'ont pas encore pu reprendre le format «

avant la fin du mois de juin ; soit le contexte sanitaire ne permettait pas la tenue d'un second tour avant fin juin et nous devions, le cas échéant, prévoir l'organisation de nouvelles élections, premier et second tours, dans les communes concernées. Le 18 mai- vous le savez -, le conseil scientifique a rendu son avis. Le Président de la République, le Premier ministre et moi-même avons ensuite consulté les associations d'élus et les formations politiques. Une décision a alors été prise- une décision prudente et responsable - : celle d'organiser le second tour des élections municipales le 28 juin. Prudente et responsable », disais-je, car cette décision doit permettre de clore ces élections municipales, mais s'accompagne de prescriptions destinées à assurer la sécurité sanitaire de la campagne et des opérations de vote. S'il s'agit d'une décision responsable,

avant-hier, s'agissant du premier de ces rapports, et le conseil a une nouvelle fois estimé que, sous réserve du respect de certaines règles sanitaires, pour la campagne électorale comme pour l'organisation du scrutin, la situation épidémiologique permettait que ce second tour des élections municipales et communautaires se tienne le 28 juin

Vous l'avez compris : le Gouvernement a souhaité par avance tenir compte de telles hypothèses ; c'est le sens de l'amendement présenté à l'Assemblée nationale visant à permettre le report localisé de l'élection du fait de circonstances sanitaires Le conseil scientifique a en outre indiqué qu'il rendrait un nouveau rapport le 14 juin, c'est-à-dire deux semaines avant la date prévue du scrutin. Si, par malheur, la situation sanitaire se détériorait d'ici là, il se pourrait que nous nous devions annuler la tenue du second tour le 28 juin. Évidemment, je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas ; mais nous devons nous tenir prêts. C'est le sens même du texte que nous examinons aujourd'hui. La situation est certes,

Deux précisions me semblent importantes, toutefois. Premièrement, dans les communes de moins de 1 000 habitants où l'ensemble des conseillers municipaux n'ont pas été désignés à l'issue du premier tour, les élus du 15 mars ont été élus définitivement. L'éventuel nouveau cycle électoral ne portera donc que sur le renouvellement des sièges encore vacants, et les nouveaux élus entreront en fonction à l'issue du nouveau scrutin. J'ajoute qu'il en va de même pour les conseillers d'arrondissement et conseillers de Paris élus au premier tour. Deuxième précision,

La jurisprudence avait déjà validé la possibilité d'annulations partielles liées, par exemple, à des coulées de boue ou à des tremblements de terre.

prise pour le moment. Ce texte organise par ailleurs la continuité de la vie des institutions locales. Dans les communes où un vote resterait à organiser, le mandat des élus actuellement en place serait prolongé, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants où des conseillers municipaux restent à désigner. intercommunale (EPCI), chacun a en tête, ici plus qu'ailleurs, leur rôle central dans l'investissement comme dans l'organisation des services publics du quotidien ; ce rôle justifie qu'ils reprennent le travail, en tenant compte des élections. Le texte prévoit donc la réunion d'assemblées « mixtes » composées de nouveaux élus et d'élus dont le mandat est prolongé. Dans ces EPCI, un exécutif provisoire sera désigné jusqu'aux nouvelles élections. Troisième finalité de ce texte : permettre la clôture du cycle électoral engagé, y compris si le second tour ne pouvait pas se tenir. Ainsi, le projet de loi prévoit le remboursement des frais de campagne engagés par les listes au titre des scrutins prévus les 15 et 22 mars juin. Quatrième objectif de ce texte concernant les élections municipales : donner à chaque Française et à chaque Français l'occasion de se rendre aux urnes et d'exprimer son choix. Un certain nombre de mesures réglementaires ont déjà été prises ou vont l'être pour favoriser le recueil des procurations, pour assurer la bonne publicité des professions de foi et des affiches des candidats et pour garantir l'organisation du scrutin dans le respect des règles sanitaires. Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin encore et déposer des amendements pour autoriser les mandataires à porter non plus une, mais deux procurations au maximum.

Nous tomberons d'accord sur beaucoup d'entre elles- je pense en particulier à quelques précisions rédactionnelles bienvenues et à des dispositions qui enrichissent le texte, par exemple la prise en compte des démissions, ou encore l'extension de la « double procuration » dans les communes où l'élection serait reportée. Je veux en revanche d'ores et déjà confirmer que le Gouvernement est opposé à certaines initiatives- nous en reparlerons tout à l'heure. Notre premier désaccord concerne la faculté de porter la procuration d'un membre de sa famille dans une autre ville que celle où l'on est inscrit sur les listes électorales. Lors de l'examen de la proposition de loi défendue par le sénateur Cédric Perrin, Laurent Nunez avait déjà exprimé notre inquiétude- non pas notre opposition de fond, mais notre inquiétude -à propos d'une telle disposition, en l'absence de mesure permettant de contrôler le nombre total de procurations susceptibles d'être détenues par un même mandataire, et donc le risque de fraude qui pourrait en découler. Autre point de désaccord : le choix de la date du 1 novembre 2020 pour l'entrée en fonction des nouveaux élus là où les élections seraient reportées, date qui serait fixe, quel que soit le jour du vote. Ce choix nous interroge ; je peine à comprendre pourquoi on priverait les nouveaux élus de l'exercice de leur mandat et pourquoi l'on s'interdirait une approche au plus près des territoires, permettant l'entrée en fonction des élus dès que possible, là où ils auront pu être élus- mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi comporte deux volets. Le premier, que nous venons d'évoquer, concerne les élections municipales ; le second porte, quant à lui, sur le report nécessaire des élections consulaires. Vous le savez, ces élections auraient dû se tenir les 16 et 17 mai C'était impossible compte tenu de la situation sanitaire et des mesures de confinement mises en place dans les différents pays du monde. Aussi le scrutin avait-il été reporté au mois de juin Là encore, nous nous sommes interrogés sur notre capacité à organiser ce scrutin, en nous fondant sur l'avis du conseil scientifique. Il apparaît clairement que l'épidémie n'est pas encore maîtrisée dans le monde, et qu'il serait impossible d'organiser ce vote dans de bonnes et égales conditions d'ici la fin du mois. On constate même, sur certains continents, sur certains continents, une aggravation de la situation. Le projet de loi prévoit donc de reporter ce scrutin au mois de mai 2021. Cette date nous donnerait plus de latitude quant à l'évolution mondiale de l'épidémie et permettrait de surcroît de ne pas avoir à décaler

c'est une démarche inhabituelle qu'a engagée le Gouvernement, dans des circonstances qui le sont tout Tout compte fait, je ne lui reprocherai pas d'avoir convoqué les électeurs pour le 28 juin le jour même où il décidait, en conseil des ministres, de saisir le Parlement d'un projet de loi portant annulation des mêmes élections. Je pourrais le faire, car c'est étonnant ... En revanche, je lui reprocherai de nous faire débattre de ce texte alors qu'il avait tout le temps, précisément, d'attendre, étant rompu à l'exercice de faire délibérer le Parlement sous trois jours quand les circonstances le justifient, et alors même que nous l'acceptons dans ce

en fonction de circonstances hypothétiques, alors qu'il pourrait fort bien intervenir utilement si ces circonstances se réalisaient. Le mois dernier, nous avons compté un million de chômeurs de plus à cause de la crise provoquée par cette terrible épidémie. Les difficultés des entreprises induisent des difficultés sociales majeures, et nous devrions, nous, consacrer beaucoup de temps à reporter des élections municipales dont tout indique qu'elles vont vraiment se tenir le 28 juin le 28 juin ? Garder au frais, au cas où, un texte adopté par le conseil des ministres, nul ne vous en aurait fait le reproche. Mais que vous ayez fait légiférer l'Assemblée nationale qui, sans mot dire,

Je vous suggère, puisqu'il faudra bien que vous débranchiez ce processus législatif à un moment ou à un autre, d'accepter ce que nous allons faire.

pour qu'il ne traite pas de questions virtuelles, mais, en revanche, maintenir dans ce texte les questions dont nous sommes certains qu'il faut les trancher. C'est le cas pour l'élection des conseillers consulaires,

pour les électeurs, mais aussi pour les membres des bureaux de vote et les candidats, le déroulement du scrutin du 28 juin. Il est assez difficile de prendre des mesures pour sécuriser ce scrutin et en même temps de l'annuler, évidemment par conséquent vous proposer d'amplifier le régime des procurations- nous discuterons des procurations données à des membres de la famille ; j'ai compris que vous étiez en désaccord avec nous sur ce point. C'est vraiment important : c'est un problème certain- tranchons les problèmes certains certains ! En revanche, ne créons pas de confusion dans l'esprit des élus locaux de France,

ne contribue d'ailleurs pas à motiver nos concitoyens à aller voter le 28 juin. Que feront-ils à force d'entendre dire que cette élection va être annulée et de voir qu'une institution réputée sérieuse- j'espère qu'elle l'est ! -, le Parlement, adopte des dispositions pour annuler un scrutin pour lequel les électeurs sont convoqués

En tout cas, je suis heureux que le président du Sénat ait écrit au Premier ministre, la semaine dernière, pour qu'au moins pendant ce débat nous ayons à notre du conseil scientifique. Il nous est parvenu avant-hier soir ; c'est très bien : nous avons pu le prendre en compte. Il n'ajoute rien au précédent avis. Et le Premier ministre, qui a satisfait avec beaucoup d'empressement à la demande du président du Sénat, est allé au-delà de nos attentes en demandant un deuxième avis pour le 14 juin.

au Sénat de faire disparaître de ce projet de loi, puisque ces dispositions sont purement virtuelles. J'ai remarqué que l'Assemblée nationale avait tout de même compris qu'il était difficile d'exposer le Président de la République à la promulgation d'une loi qui aurait été adoptée en termes identiques par les deux assemblées et qui, alors, devrait s'appliquer bien que le décret de convocation des électeurs soit resté en vigueur. Eh oui, c'est vrai : il y a un grand danger à mettre le Président de la République dans l'embarras

C'est une des raisons pour lesquelles, de toute façon, il ne fallait pas que le Sénat adopte conforme le texte de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale a compris les choses ; elle a donc dit- je restitue

posé la question de la conformité à la Constitution d'une telle démarche. Et a surgi dans ma mémoire la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1986.

supprimerait de ce texte toutes les dispositions relatives au report des élections municipales. Avec un maximum de bienveillance pour le Gouvernement, cette dernière voie est celle sur laquelle j'ai engagé la commission des lois. Avec un peu de chance, monsieur le ministre,

dont nous aurons décidé ici, ce que je préférerais, parce que cela réglerait le problème des procurations et de la sécurité du vote du 28 juin et celui des délégués consulaires, ces deux problèmes étant, eux, certains et essentiels.

le déconfinement marque une étape importante dans la lutte contre l'épidémie ; avec lui, c'est aussi la vie démocratique et électorale qui reprend son cours. Ce mouvement Ce mouvement a été engagé dès le 13 mai, avec l'installation des conseils municipaux complets de 30 000 communes. Toutefois, à ce jour, 5 000 communes sont encore dans l'attente d'un deuxième tour. C'est la dernière étape avant le retour à une vie démocratique normale, celle-ci s'étant trouvée largement bouleversée par cette crise. Cette vie démocratique ne s'est pourtant pas interrompue, grâce au travail et à l'engagement quotidiens des maires et de tous les élus locaux. Les maires ont su, tout au long de cette crise, illustrer leur rôle d'élus de proximité. Chacun d'entre nous, par nos échanges et nos contacts permanents avec eux, peut en témoigner : ils n'ont jamais ménagé leurs efforts. Les maires ont indéniablement su répondre à l'urgence. Ils ont partout tenu leur rôle de garants du lien social auprès de leurs administrés, quand ces derniers avaient une question à poser sur le confinement, et notamment auprès des personnes les plus vulnérables, les personnes âgées et les personnes isolées. Ils ont su aussi organiser la reprise de la vie scolaire, dans des conditions souvent difficiles. Nous savons que les collectivités territoriales, au premier rang desquelles le bloc communal, seront les maillons essentiels de la reprise, par la commande publique, par l'investissement, par le redémarrage des chantiers, par tous ces leviers que peuvent actionner les communes et leurs EPCI. Pour toutes ces raisons, démocratiques, sociales, économiques, il est primordial de prévoir la possibilité d'un report encadré du deuxième tour des élections municipales, même circonscrit à quelques communes, et d'en anticiper les conséquences, si les conditions sanitaires ne permettaient finalement pas sa tenue. L'obligation pour le Gouvernement de consulter le conseil scientifique, ajoutée par nos collègues députés, est une mesure de bon sens, mais aussi un gage de sérieux et de crédibilité. le message suivant : « Cette décision, qui consiste à vous demander de prendre toute votre part dans notre vie démocratique, est mûrement réfléchie et pesée ». Ce sérieux, nous le devons à tous les Français comme à nos candidats et à nos élus. Nous le devons à tous ceux qui, durant ces trois derniers mois, ont accepté de restreindre leurs libertés au nom de l'intérêt général. C'est ce sens de l'intérêt général dont ont fait preuve les Français qui doit nous inspirer et doit guider nos choix. Ce projet de loi nous permet de prévoir et d'encadrer un report localisé du scrutin. Il ne traduit aucune forme de pessimisme, mais témoigne bien plutôt du sérieux dont nous souhaitons et devons collectivement faire preuve. Ce sérieux, c'est celui de l'impérieuse nécessité d'envisager tous les scénarios possibles, afin de ne mettre personne en danger : voter ne doit pas se faire aux dépens de la santé des Français- le scénario de Ce sérieux, c'est également celui que nous devons à l'ensemble de nos élus. Nous le devons à nos actuels élus locaux- je pense notamment à tous ces maires sortants qui ne se sont pas représentés et qui voient leur mandat prolongé depuis le 15 mars dernier, ceux-là mêmes qui, alors qu'ils avaient laissé la place à d'autres, ont mis leur temps et leur énergie au service de leurs concitoyens, tout au long de la crise, sans jamais faillir. à nos futurs élus, nous leur devons une situation clarifiée, et un vote se déroulant dans des conditions sanitaires optimales. Ce projet de loi naît- je l'ai dit -d'un constat partagé : celui de la nécessité d'anticiper une hypothèse de dégradation de la situation sanitaire.

Oui ! Je souhaite leur répondre que, si cela peut sembler original, il n'en reste pas moins que c'est une nécessité. Celle de l'anticipation, celle de la précaution à l'égard de tous les Français. Le Gouvernement nous présente donc un projet de loi complet, utilement enrichi par nos collègues députés, un texte à la hauteur des enjeux sanitaires, démocratiques et politiques. a fait le choix de supprimer les dispositions éventuelles qu'il prévoyait pour lui préférer des mesures certaines, qui répondent de façon pratique aux multiples complexités qui nous attendent. Mes chers collègues, les apports de l'article 5 collègues, les apports de l'article 5 de ce texte sont véritables, puisqu'ils permettent de prévoir l'annulation et le report par décret en conseil des ministres du scrutin uniquement dans certaines communes dans lesquelles une recrudescence de l'épidémie adviendrait. C'est là une disposition tout à fait adaptée à la réalité mouvante des phénomènes de clusters. Je veux également dire notre satisfaction devant l'article 4 de ce projet de loi, qui vise à reporter les élections consulaires au mois de mai 2021. Ces dispositions répondent à l'attente légitime de tous les candidats aux élections de délégués et de conseillers consulaires, et plus largement de l'ensemble de nos compatriotes établis à l'étranger. C'est un choix prudent et une date raisonnable. Nous soutiendrons aussi les dispositions précautionneuses qui nous permettent d'anticiper les corolaires d'une possible annulation du scrutin dans certaines communes. Les règles de campagne et de financement pourraient ainsi être adaptées dans les communes où le scrutin serait annulé. Le texte dont nous débattons aujourd'hui comprend également de nombreuses mesures pour un fonctionnement allégé des collectivités territoriales. Je pense, par exemple, à l'extension de l'assouplissement des règles de quorum, à la possibilité de tenir les réunions de l'assemblée délibérante par visioconférence ou encore à celle offerte aux conseils municipaux et communautaires de se réunir en tout lieu. Enfin, nous soutiendrons ce texte, car le Gouvernement a su tenir de nouveau son engagement de ne jamais oublier les territoires ultramarins. L'article 6 vise ainsi à satisfaire la demande de souplesse et de compréhension pour adapter le régime électoral à la réalité insulaire de Polynésie française. Chers collègues,

puisqu'une grande partie des dispositions de ce texte n'avaient pas vocation à être appliquées si le second tour a bien lieu le 28 juin, ce qui semble être en bonne voie, d'où notre approbation quant aux suppressions décidées par la commission des lois.

Alors que le Conseil constitutionnel se prononcera lundi prochain sur la constitutionnalité de la tenue des élections municipales, le Gouvernement poursuit avec ce

L'ajout, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, d'un article visant à permettre d'annuler partiellement le second tour dans les communes où la circulation du virus serait toujours trop intense pour que le scrutin puisse se tenir en est l'exemple, et nous regrettons que la commission ait conservé cet article. de même de l'oubli de recueillir l'avis du Congrès de Nouvelle-Calédonie sur certaines dispositions concernant ce territoire, qui a fait décaler l'adoption du texte. Les conditions d'examen étaient déjà contestables la semaine dernière, mais ce report ce report les a rendues d'autant plus compliquées, monsieur le ministre. Nous ne pouvons accepter de travailler de cette façon. L'exécutif veut assumer son choix du maintien du second tour en juin, mais dans son désir d'anticipation le Gouvernement manque de cohérence et perd du monde sur la route de la démocratie Pour revenir sur l'article que j'appelle « foyers épidémiques », pour ne pas reprendre le mot clusters, imaginons qu'il y ait des communes où l'on annule le second tour alors que celui-ci est maintenu pour le reste du territoire.

deux nouveaux tours d'ici octobre 2020 pour les communes identifiées « foyers de transmission », sans parler des élections sénatoriales dont nous discuterons aussi dans un contexte incertain dans quelques jours et sur lesquelles une annulation même partielle aurait un impact.

Le feu plutôt orange du comité de scientifiques devrait passer au vert dans quelques jours, et tous les élus et candidats pourront enfin sortir de cet étrange entre-deux. La commission des lois estime avoir « purgé » le projet de loi des dispositions « virtuelles », mais « virtuelles », mais le maintien de l'article 5 implique le maintien de toutes les dispositions anticipant une annulation du second tour qui ne devraient pas être appliquées. Il en va ainsi du choix de fixer la prolongation des mandats et des entrées en fonction alors que de telles dates ne relèvent pas de notre compétence : elles dépendent d'un hypothétique futur sur lequel nous n'avons pas la main. Les autres dispositions qui ont vocation à s'appliquer et qui ont été complétées en commission sont majoritairement de bon sens. Elles visent à favoriser la participation et à faciliter la vie démocratique locale, qui doit être conciliée avec les exigences sanitaires et les conséquences du report du second tour. Néanmoins, nous nous opposons à ce qu'une procuration puisse être établie entre un mandant et un mandataire résidant dans des communes différentes, même s'ils ont un lien de filiation. La participation citoyenne ne doit pas reposer sur de telles bases. En ce qui concerne les Français de l'étranger, qui ne pourront élire leurs conseillers consulaires et délégués consulaires au regard de l'hétérogénéité des situations à travers le monde, nous sommes favorables au report de ces élections en mai 2021. Sur la forme, nous nous rallions à l'avis du Conseil d'État en déplorant la méthode utilisée par le Gouvernement et reprise par la commission des lois pour rédiger ce texte en décortiquant la loi d'urgence du 23 mars et les ordonnances passées, plutôt que de rassembler les nouvelles dispositions dans un texte autonome.

sur ce texte, en cohérence avec notre position quant à la gestion gouvernementale des élections municipales. Selon la tournure de nos débats, nous nous réservons la possibilité de voter contre ce texte, notamment si la généralisation du vote par correspondance était adoptée.

Capus. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 5 juin dernier, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, déclarait que l'épidémie semblait être sous contrôle. Avec un millier de nouveaux cas par jour, comparés aux 80 000 contaminations quotidiennes du début du mois de mars, notre pays a de bonnes chances de vaincre la pandémie.

de prévoir les conditions de l'annulation des élections municipales pour le cas où le contexte sanitaire ne permettrait pas la tenue du second tour le 28 juin prochain. Comme l'a parfaitement souligné le président Bas, il y a quelque chose de paradoxal à discuter d'un texte en espérant qu'il ne trouvera pas à s'appliquer.

Le vrai courage, c'est la prudence », disait Euripide avec raison. Durant les derniers mois, nous avons entendu bon nombre de voix s'élever pour affirmer avec certitude ce qui aurait dû être fait pour éviter la crise. Certains ont aussi chanté les louanges de remèdes miracles, reconnus par tous, et surtout par ceux qui les proposaient ! Au-delà des théories du complot, la réalité nous incite à la prudence et à l'endurance. La résolution de la crise viendra plus certainement d'un travail et d'un effort dans la durée que de coups d'éclat. La pandémie a fortement perturbé le fonctionnement de notre pays. Après la grave crise sanitaire qui, nous l'espérons, se trouve déjà derrière nous, nous allons devoir faire face à une crise économique historique. Une fois de plus, les maires ont montré qu'ils sont des figures incontournables de la gestion de crise dans nos territoires. Ils ont tenté sans relâche de répondre aux attentes de leurs administrés dans des conditions particulièrement dégradées. Beaucoup d'entre eux ont pris des mesures permettant de ralentir la propagation du virus, notamment en assurant une distribution de masques à nos concitoyens. Le virus a touché tous les aspects de l'activité de notre société. Les processus électoraux n'ont pas été épargnés. Alors que l'action de nos collectivités est plus nécessaire que jamais, près de 5 000 communes et 16,5 millions d'électeurs sont à ce jour dans l'attente d'un second tour. Tout en veillant à préserver la santé des votants et des organisateurs du scrutin, nous pensons que la tenue du second tour est à cet égard impérative pour permettre aux équipes municipales d'agir avec une légitimité pleine et entière. Dans cette optique, nous saluons l'assouplissement du régime de procuration de vote. Beaucoup de personnes fragiles, ou en contact avec des personnes fragiles, ne sont pas allées voter le 15 mars dernier. La participation s'en était ressentie. Nous devons créer les conditions d'une participation plus large pour les prochaines élections. Le conseil scientifique a indiqué avant-hier, ce qu'il devrait confirmer le 14 juin prochain, que les circonstances sanitaires du second tour sont bien meilleures que celles du premier Le virus semble être sensible aux saisons : c'est heureux pour nous à l'approche de l'été, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle contamination ou même d'une nouvelle maladie. Il nous faut donc anticiper les situations dans lesquelles le vote classique peut être problématique. Pour cela, nous pensons que le système de la procuration de vote pourrait être revu afin de mieux l'adapter aux contextes de crises. Tel est le sens d'un amendement que j'ai déposé : il vise à permettre au mandataire, et non plus seulement au mandant, de faire les démarches

D'autres pistes, souvent évoquées, sont celles du vote électronique ou encore du vote par correspondance. La commission a ajouté à cet égard la possibilité du vote par correspondance sur support papier pour les conseillers représentant les Français de l'étranger. C'est une bonne chose. Plus généralement, il conviendrait de lancer une étude approfondie sur les différents types de vote afin de déterminer leur pertinence et leur fiabilité. En effet, si l'épidémie recule, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle dégradation des conditions sanitaires. À ce sujet, nous remarquons que le texte vise à prévoir avec sagesse la possibilité d'annuler le second tour dans des communes qui seraient touchées par une résurgence du virus. Ce risque n'est pas à exclure et nous voyons dans cette mesure une prudente précaution. En plus du vote, c'est l'ensemble des conditions du scrutin, notamment la campagne électorale, qu'il conviendrait d'ajuster aux contextes de crise. Les dispositions contenues dans ce texte nous apparaissent nécessaires. Nous espérons et nous croyons que le recul de l'épidémie permettra de ne pas faire application de bon nombre d'entre elles.

l'intitulé officiel du projet de loi que nous examinons aujourd'hui est très long, mais il pourrait être assez aisément simplifié : ce serait alors un projet de loi « au cas où » : au cas où la situation sanitaire ne permettrait pas l'organisation du second tour des élections municipales le 28 juin prochain Mission assez inédite pour le législateur auquel le Gouvernement propose d'adopter des dispositions dont il ne sait pas si elles ont réellement une utilité et si elles entreront en vigueur un jour. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui résulte, bien sûr, de la crise sanitaire sans précédent qui touche notre pays et l'ensemble du monde depuis plusieurs mois. Mais cette situation découle également des choix que nous avons faits, des choix du Gouvernement en réalité : fallait-il organiser le premier tour d'une élection sans savoir si nous aurions la capacité d'organiser le second ? Fallait-il même organiser une élection alors que la pandémie était déjà là et que nous étions à la veille d'un confinement généralisé ? Je n'ai nullement l'intention d'alimenter des polémiques, mais une chose est certaine : depuis la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, nous avons examiné de très nombreuses et très complexes dispositions en matière électorale et d'organisation des collectivités territoriales dont nous aurions pu faire l'économie si nous avions décidé d'organiser ces élections une fois la pandémie maîtrisée. Et je ne parle pas du contentieux électoral qui, hélas ! ne manquera pas d'être multiplié par les différents éléments que je viens de rappeler ... Le texte transmis au Sénat, adopté par l'Assemblée nationale lundi après-midi, prévoyait donc ce qui se serait passé si les conditions sanitaires n'avaient pas été réunies pour organiser un second tour des municipales le 28 juin prochain. Notre président-rapporteur de la commission des lois a brillamment exposé la stratégie qui a guidé les travaux la stratégie qui a guidé les travaux de la commission hier matin : nous ne pouvions pas sérieusement continuer à faire du droit virtuel, du droit « au cas où ». Nous avons donc considéré que, à l'exception quelques zones ciblées où la situation sanitaire serait incompatible avec un second tour- les fameux clusters -, le scrutin aurait bien lieu le 28 juin. Notre groupe tient à saluer le travail effectué par la commission. Une fois n'est pas coutume, elle a dû examiner ce projet de loi dans des conditions de temps extrêmement strictes qui, soyons honnêtes, ne permettent pas au législateur d'exercer sereinement sa mission, d'autant que cette méthode de travail ne se justifie par aucune contrainte calendaire réelle. Pour reprendre les mots de notre rapporteur, « elle ajoute inutilement de la confusion non seulement pour le Parlement, mais également pour les candidats et les électeurs appelés aux urnes dans une période déjà très incertaine Par ailleurs, on peut s'interroger sur le choix du Gouvernement consistant à décorréler l'examen de ce projet de loi du projet de loi organique que nous avons examiné ce matin en commission, et qui est fondamentalement lié au texte que nous Cela a été rappelé, notre commission des lois a donc assez largement remodelé le texte transmis par l'Assemblée nationale en tenant compte des dernières conclusions du comité de scientifiques sur le contexte sanitaire, rendues lundi soir.

Mais chacun a bien compris que nous devions continuer à nous protéger contre le virus qui, lui, n'a pas disparu. Il fallait donc que nos concitoyens les plus fragiles puissent exercer leur droit de vote sans risquer d'être inutilement exposés à un risque de contamination. Ce texte était donc l'occasion de reprendre un certain nombre de dispositions votées par la Haute Assemblée la semaine dernière tendant à faciliter, notamment, le recours aux procurations. J'espère que les apports du Sénat sur ce point seront repris par nos collègues députés, car il s'agit de mesures de bon sens, qui n'ont qu'un seul objectif : faire en sorte que le maximum de nos compatriotes puisse voter tout en leur assurant le meilleur niveau de sécurité sanitaire. Il est important de les rassurer sur ce point. Je me félicite aussi que le texte de la commission ait intégré plusieurs amendements déposés par des membres de mon groupe, notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales. Il était, par exemple, nécessaire d'adapter le calendrier de renouvellement de certaines instances comme les comités Le texte voté en commission vise à prévoir que le comité des syndicats mixtes fermés pourra tenir sa réunion d'installation jusqu'au vendredi 25 septembre, ce qui permettra d'éviter que ces réunions n'interviennent en plein mois d'août un mot enfin sur le sujet qui devient pratiquement le coeur du texte, à savoir l'annulation des élections consulaires. Notre commission a intégré plusieurs dispositions, dont certaines avaient déjà été adoptées par le Sénat dans le cadre de l'examen de récentes propositions de loi, afin d'assurer le bon déroulement des élections consulaires, mais aussi visant à mieux reconnaître l'engagement des élus représentant les Français de l'étranger. Nous avons ainsi fixé une date certaine- en mai 2021 -pour les prochaines élections consulaires et autorisé le vote par correspondance sur support papier, dans des conditions garantissant la sincérité et le secret du vote. Nous avons également amélioré les conditions d'exercice du mandat des conseillers des Français de l'étranger, notamment pour mieux concilier leurs fonctions électives et leur vie professionnelle : reconnaissance des acquis de l'expérience, autorisations d'absence, prise en charge des frais de transport, etc. Reste la délicate question de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France dont le report est prévu dans le projet de loi organique que j'évoquais précédemment et que le Gouvernement n'a pas souhaité nous faire examiner aujourd'hui C'est bien dommage, car, naturellement, la question du report des élections consulaires est profondément et intimement liée à celle des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Mais je n'en dis pas plus sur ce thème aujourd'hui, car c'est la semaine prochaine que le Sénat devra délibérer sur cette question. Je tiens une fois encore à saluer, mes chers collègues, le travail réalisé par le président Philippe Bas. Il nous a permis à la fois d'évacuer de ce projet de loi son caractère hypothétique et d'enrichir le texte en y intégrant des dispositions auxquelles Sénat avait marqué son attachement

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées le 15 mars dernier pour rendre possible le premier tour des élections municipales dans des circonstances si particulières

que nous pouvons faire vivre la politique de manière concrète. Dans la crise sanitaire, le rôle des collectivités locales a été essentiel.

la convocation des électeurs le 15 mars et la déclaration du Premier ministre du 14 mars, on peut dire que, au moins au début de la pandémie, l'improvisation de l'État central n'avançait pas masquée Depuis, les choses ont un peu évolué. Quoi qu'il en soit, nous avons eu besoin des collectivités locales au moment de cette crise et il faudra réfléchir à l'organisation de notre État à la suite de cela. Le contexte actuel

ce qui fait également peser un certain nombre d'incertitudes sur l'ensemble du scrutin. Enfin, le rapport du conseil scientifique du 8 mai dernier, même s'il signale une évolution globalement positive, note qu'il existe des difficultés spécifiques à Mayotte et en Guyane. Or la Guyane, comme les Français de l'étranger, doit procéder à un renouvellement sénatorial en septembre. C'est donc en tenant compte de ces nombreuses incertitudes que nous devons nous décider aujourd'hui sur le projet de loi qui nous est présenté.

nous la vivons depuis trois mois, nous savons maintenant ce que c'est ! -, ceux qui vivent également une tragédie sans précédent dans certains pays d'Amérique latine, en Amérique du Nord,

L'apport principal de notre rapporteur et de notre commission est de proposer de n'inscrire dans la loi que ce qui est certain. Cette clarification a engendré d'ailleurs dans la nuit une autre clarification,

Enfin, concernant les élections consulaires, notre commission considère- et c'est heureux -qu'il convient de respecter à la fois les électeurs et les candidats qui font vivre la démocratie locale, en fixant définitivement une date pour les élections de 2021. Ces élections ont déjà été reportées une fois de fin mai à fin juin. Il conviendra maintenant de dire

chers collègues, il est tout à fait singulier de débattre en cet instant d'un texte dont, selon toute vraisemblance, certaines dispositions initiales ne s'appliqueront jamais. Si, comme le disait Pierre Mendès France, « gouverner c'est prévoir et s'il fallait bien prévoir l'hypothèse d'un report de ces élections, compte tenu des délais constitutionnels et du nécessaire respect du Parlement, la méthode proposée ne cesse de nous étonner. Quoi qu'il en soit, sur la forme, je me réjouis que nous puissions prochainement tourner la page de ces élections municipales. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est la Bigourdane que je suis qui vous le dis ! En effet, il aurait été intenable de continuer pendant presque un an avec ce mélange d'élus sortants et de nouveaux élus qui, dans nos territoires, serait venu mettre à mal l'équilibre de nombreuses intercommunalités- elles n'ont pas besoin de cela ! -, sur lesquelles il faudra compter pour relancer notre économie.

se sont acquittés jusqu'au bout de leur mandat afin de garantir le bien-être, la sécurité et l'intérêt général de leurs administrés durant cette période de crise. C'est aussi cela, le sens du service public Pour en revenir au texte, je tiens à saluer le choix de notre commission et de son rapporteur de ne pas légiférer sur de l'hypothétique ; je pense au report des élections municipales, mais aussi au renouvellement de nos collègues sénateurs de la deuxième série. Comme cela a été rappelé, si nous devions reporter ce second tour, rien ne s'opposerait à l'adoption d'une nouvelle loi de report, qui cette fois se concentrerait non pas sur des hypothèses, mais bien sur des faits et une situation qui se serait passablement dégradée. Sur le scrutin qui nous attend le 28 juin, il y a fort à parier que nous ne puissions manifestement pas garantir aux citoyens d'avoir deux procurations, et nous le regrettons. Après la faible participation du premier tour, il aurait été de bonne politique de faciliter le recours aux procurations, dans le prolongement de nos débats de la semaine dernière. Ce scrutin pourra sans doute se tenir, mais il faut garder en tête que le virus est toujours là, et beaucoup de personnes fragiles ou même atteintes par le virus n'iront pas voter. Pour ce qui concerne les débats sur le vote par correspondance, il aurait été, à mon sens, trop complexe oeuvre ce dispositif dans des délais aussi brefs, ce qui aurait soulevé au passage trop d'incertitudes et d'insécurité juridique. Sur l'installation des comités syndicaux, le calendrier des délibérations indemnitaires ou encore les délais de convocation des assemblées communautaires, les membres du RDSE souscrivent pleinement aux modifications proposées par la commission, qui viennent clarifier la situation. La principale inquiétude qui demeure est celle pesant sur le renouvellement de nos collègues représentant les Français de l'étranger, du fait du report de l'élection des conseils consulaires. Celui-ci était inévitable et nous conduit à proroger le mandat des conseillers sortants jusqu'à la fixation de nouvelles élections. Si la date de mai 2021 doit pouvoir être retenue, nous ne sommes pas à l'abri de difficultés, car nous ne pouvons prévoir l'évolution de l'épidémie dans le monde. Le recours au vote par correspondance ne suscite aucune opposition de notre part, compte tenu du caractère très particulier de ce scrutin. Vous l'aurez compris, le RDSE approuvera ce texte. Délesté, grâce au travail du Sénat et de notre rapporteur, de ses dispositions hypothétiques, il permettra que ces scrutins se déroulent de la meilleure des manières. La parole présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au début de la séance, nous discutions d'un projet de loi « relatif à diverses dispositions ». Nous poursuivons maintenant avec un texte qui, dans la version au titre fort long que nous avait transmise l'Assemblée nationale, portait essentiellement sur des dispositions En ces temps de crise sanitaire exceptionnelle, nous avons désormais, malheureusement, pris l'habitude de consentir à des mesures tout aussi exceptionnelles, souvent dans l'urgence, avec conscience des enjeux, prudence et discernement. C'est pourquoi ce projet de loi ne surprend guère. Il vise, de prime abord, à annuler le second tour des élections municipales de 2020, ainsi qu'à reporter les élections consulaires, alors même que, il y a une semaine à peine, nous votions une proposition de loi de notre collègue Cédric Perrin portant sur ces élections. À ce moment-là, le Gouvernement nous indiquait que certaines mesures de facilitation de l'organisation du vote prévues dans la proposition de loi trouveraient leur place dans ce projet de loi annulant les élections. Celui-ci a ainsi été proclamé « vecteur législatif approprié » pour parler de leur bon déroulement. Certains députés de la majorité ont ainsi repris l'idée de doubles procurations, présente dans la proposition de loi du Sénat, et l'ont inscrite dans un texte qui, en même temps, établit un régime d'annulation hypothétique de ces mêmes élections. Vous avouerez que c'est un peu surréaliste ! Pourquoi un régime hypothétique ? Parce qu'il implique que le second tour pourrait être annulé par simple décret si la situation sanitaire à la veille du scrutin l'imposait. Pourquoi pas ? Une dégradation subite de la situation sanitaire, même si elle est peu probable, n'est pas impossible. Cependant, légiférer de la sorte présente des difficultés. Dans son avis, le Conseil d'État relève avec sa prudence coutumière l'étrangeté d'une situation dans laquelle il est appelé à se prononcer sur des dispositions, sans que les conditions requises pour décider de leur mise en oeuvre soient réunies. Les parlementaires sont désormais placés face à la même situation, et nous sommes nombreux à ne pas apprécier cette manière de procéder. Notre commission, sur l'initiative de son président et rapporteur Philippe Bas, s'est efforcée de clarifier les choses : « Le Parlement n'a pas vocation à trancher des questions hypothétiques, cela non seulement parce qu'il y a une infinité de situations possibles, mais aussi et surtout en raison des fragilités constitutionnelles d'une pareille démarche. » En effet, le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné par le passé des cas dans lesquels le législateur laissait à l'exécutif le choix de l'entrée en vigueur ou non de dispositions législatives. Par contraste, le dispositif de l'article 5 soulève moins d'interrogations. Certes, il permettra au Gouvernement d'annuler le scrutin dans les communes les plus touchées par l'épidémie.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a supprimé les dispositions virtuelles du texte, se plaçant ainsi dans la continuité de Montesquieu lorsqu'il écrivait : « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Elle a oeuvré pour renforcer ce qui est nécessaire et a introduit des garanties importantes pour le bon déroulement des élections du 28 juin, notamment à partir de mesures déjà présentes dans la proposition de loi sénatoriale tendant à sécuriser l'établissement des procurations Parmi ces garanties, il y a la possibilité d'établir une procuration en faveur d'un proche, des aménagements pour cette mise en place au bénéfice d'électeurs vulnérables, ou encore la garantie que des équipements de protection soient mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Outre ce qui concerne directement les élections municipales, le projet de loi comprend désormais un certain nombre d'autres éléments. Il s'agit, par exemple, de dispositions visant à prolonger des aménagements très concrets au fonctionnement normal des collectivités durant les mois à venir. Ceux-ci contribueront à concilier sécurité sanitaire et bon déroulement de la vie des institutions locales. D'autres éléments permettront de rétablir des délais plus en phase avec le droit commun pour le contentieux électoral du scrutin du 15 mars, ou encore d'ajuster certaines dispositions relatives aux grands électeurs en Polynésie. Le troisième volet de ce texte concerne la représentation des Français de l'étranger. La situation sanitaire globale a rendu le report des élections consulaires inévitable, et nous en prenons acte par la fixation d'une date certaine en mai 2021. Toujours dans la lignée de ce qui a été voté, nous proposons aussi le vote par correspondance sur support papier qui, associé à des garanties procédurales, nous semble approprié en ces temps d'obstacles à la mobilité. Je tiens à signaler ici la reprise, sur l'initiative de nos collègues représentants des Français de l'étranger, d'un certain nombre d'avancées issues de plusieurs textes que notre assemblée a déjà votés, pour certaines pas plus tard que le 19 mai dernier. la proximité de l'action publique, mais ont vu leur calendrier remis en cause par le report des élections consulaires. Par exemple, nous permettrons à des élus de présider les conseils consulaires dès octobre 2020, répondant ainsi à une demande ancienne. En somme, grâce à l'adoption en commission d'amendements relatifs à ces sujets, le projet de loi permettra une entrée en vigueur rapide et effective de ce qui a déjà été promulgué, et donnera de nombreuses autres garanties aux représentants des Français de l'étranger. Pour conclure, c'est à raison que la commission des lois a recentré le texte sur des mesures nécessaires à l'organisation des élections municipales. Non pas qu'il ne faille pas être prêt à toute éventualité ; nous avons récemment démontré à cet égard que nous étions capables de travailler dans des conditions de temps très contraintes, alors que c'était réellement nécessaire. Mais il nous semble peu judicieux de recourir à des lois virtuelles il nous semble peu judicieux de recourir à des lois virtuelles pour parer à toute éventualité. Au contraire, nous préférons être proactifs pragmatiques sur des sujets réalistes, tels que l'organisation du second tour des élections municipales ou la représentation des Français de l'étranger. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains approuve le travail réalisé en commission et sera favorable à cette version modifiée du projet de loi. La parole est à M. le ministre.

tour des élections municipales. Le Sénat se doit de défendre les collectivités territoriales d'une manière générale. Or les conditions d'exercice de cette rencontre essentielle entre le citoyen

les clignotants sont désormais au vert sur l'ensemble du territoire national ou presque. Il est grand temps que nous refermions cette période électorale d'un type tout à fait particulier. Il faut s'en tenir à la règle démocratique habituelle et ne pas tirer

le rapporteur reprend le rôle du Gouvernement en proposant des dispositions qui ne s'appliqueront pas, et le Gouvernement fait preuve de réalisme ... On devrait pouvoir converger

vous vous surpassez ! Vous nous dites que cet article est utile parce qu'il est utile. Or il est évident qu'il est inutile, puisque le rapport sera produit le 14 juin

de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, tout en prévoyant que chaque candidat ou représentant des candidats doit désigner une personne qui sera présente. Cela me paraît bien ! Je vous recommande donc, mes chers collègues, de ne pas suivre le Gouvernement, qui veut vider d'une partie de sa substance

C'est un frein, car la personne qui souhaite donner procuration n'a pas toujours le courage, l'envie, l'opportunité ou la possibilité physique d'aller établir elle-même sa procuration. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement, qui tend à prévoir que le mandant

? Nous avons fait le même diagnostic et nous voulons traiter cette situation, mais nous préférons imposer à un agent assermenté le déplacement au domicile de la personne vulnérable, plutôt que permettre à un mandataire putatif de faire les démarches et d'aller ensuite au domicile du mandant. Pourquoi ? Parce qu'il semble que cette option-ci présente moins de garanties de vue du risque de fraude. Je le sais bien, on doit partir d'un postulat de confiance à l'égard des Français qui vont se dévouer pour un proche ou pour un membre de leur famille, mais il n'y a pas que des gens de confiance ... C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, en vous indiquant que ce que nous avons prévu me paraît

de ma circonscription qui m'a posé cette question et qui m'a alerté sur cette difficulté. Je crois beaucoup à la confiance, à la responsabilité, et faire un faux me paraît extrêmement grave. En Maine-et-Loire, je n'imagine même pas que l'on puisse

à un risque : l'électeur ne se déplace pas au bureau de vote, on ne vérifie pas sa carte d'identité et il ne passe pas par l'isoloir. Donc, évidemment, c'est un système moins sûr que le vote à l'urne ... Cela dit, quelle part de risque acceptons-nous ? Une part très faible. Quand il s'agit d'un membre de la famille- le fils, la fille, le frère, la soeur -, il est facile de prouver, avec une fiche familiale d'état civil et sa carte d'identité, l'existence de ce lien de parenté.

aux présidents des bureaux de vote de s'assurer des choses du mieux qu'ils le pourront. Empêcher, au nom de déviations marginales possibles, le le fils d'une vieille dame de voter pour celle-ci, alors qu'il n'habite pas dans la même commune et n'y est pas électeur, me paraît là aussi excessif. Il faut trouver un bon équilibre. Je ne dis pas que notre solution est parfaite, mais je la préfère à la vôtre.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, Il n'en a déposé qu'un, puisque le vote par correspondance, dont il est question ici, ne pourrait pas matériellement être mis en oeuvre pour le 28 juin

Pour cela, il fallait simplement que la proposition de loi du Sénat fasse l'objet d'une procédure accélérée, soit adoptée par l'Assemblée nationale et qu'une commission mixte paritaire soit réunie ; alors, nous aurions eu le vote par correspondance Le Gouvernement est cohérent, il n'en veut pas et, par conséquent, il n'a pas facilité l'adoption de ce texte sénatorial. Pourtant, nous avons eu quelque

on redéclenche l'état d'urgence, alors on aura eu le temps de se préparer au vote par correspondance et, au travers de votre amendement, vous voulez que l'on ne puisse plus nous opposer notre impréparation. Simplement, vous indiquez, dans la rédaction du dispositif, que c'est pour l'hypothèse où l'état d'urgence serait de nouveau déclaré, mais, je dois vous le rappeler, dans la loi du 23 mars dernier, nous avons décidé que cet état d'urgence ne pourrait être mis en oeuvre par le Gouvernement que jusqu'au 30 mars de l'année 2021.

au nom de Charles Guené. Pour les élections des intercommunalités, notamment de toute l'équipe dirigeante et du président,

et puissent prendre rapidement des décisions, avant les congés bien mérités d'août. Cet amendement est très simple, très compréhensible et peut-être qu'il recevra un avis favorable de la commission.

qu'il faut attendre quatre semaines pour réunir le conseil, l'installer et démarrer le travail. Il s'agit d'un délai maximal, donc on n'a pas besoin d'attendre ces quatre semaines. Cela dit, il est vrai qu'il y avait un problème tout à fait particulier qui tenait au délai non pas pour la réunion, mais pour la convocation du conseil. Il faut que la convocation ait lieu, si l'on ne touche pas au délai, au moins cinq jours avant la réunion. Cela tomberait, dans bien des cas,

de procurations expire au 30 août prochain. Nous avons des raisons de penser que ces facilités de réunion pourraient encore être utiles pendant les deux premiers mois suivant la rentrée, en septembre et octobre.

la cascade de conséquences du report au 28 juin du second tour des élections municipales, il y a évidemment l'installation des conseils municipaux, des conseils intercommunaux et des conseils syndicaux- syndics communaux et intercommunaux.

les syndicats communaux ou intercommunaux doivent, eux aussi, s'installer, voter leur budget et leurs comptes administratifs. C'est absolument intenable ! L'ordonnance du 25

Cela coïncide exactement avec le moment où les syndicats communaux et intercommunaux devront faire la même chose ; cela ne tient pas ! Il y a concomitance des deux événements.

du budget à l'automne ; il s'agit bien de l'adoption des comptes administratifs, par des élus qui seront installés et non par d'anciens élus, qui n'auront plus de légitimité, on le sait bien, dès lors que le second tour aura eu lieu. tour aura eu lieu. Quel est l'avis de la commission ? Mon cher collègue, s'il y a un problème spécifique aux syndicats mixtes, il faut faire un amendement sur les syndicats mixtes. Vous avez déposé un amendement qui reporte le vote des budgets des collectivités au 15 octobre 2020.

nous avons besoin de collectivités et d'établissements publics de coopération intercommunale directement opérationnels. J'ajoute que ces syndicats mixtes, qui pouvaient vivre sous un régime de douzièmes provisoires, en quelque sorte, avec l'accord du préfet, avaient parfaitement le droit, et l'ont toujours, d'adopter leur budget, quitte à ce que celui-ci soit modifié ensuite par les nouvelles équipes. Au fond, il ne faudrait pas que, du fait qu'ils se sont abstenus de faire ce qu'ils avaient le droit, et sans doute même le devoir, de faire, on modifie la loi pour toutes les collectivités locales, en retardant le vote du budget et en restant dans un régime intérimaire, qui n'est pas bon en ce moment ; du moins, je le crois. Je suis à votre disposition pour discuter du problème spécifique que vous venez

élections sénatoriales.

un certain nombre de mesures sur le quorum ou les procurations au sein des conseils municipaux valables jusqu'au mois d'octobre, mais aussi au fait que l'on puisse réunir le conseil municipal en dehors des lieux majestueux où il se réunit habituellement, dès lors qu'il n'y a plus de justification sanitaire.

de procéder par un scrutin ouvert, plutôt que par un scrutin secret.

document très lourd à produire. Or c'est un facteur important de transparence démocratique et financière, qui doit être considéré comme une annexe essentielle à l'acte budgétaire.

mes chers collègues, je tiens, à l'occasion, de l'examen de l'article 4, à remercier chaleureusement le président de notre commission des lois, Philippe Bas, qui est toujours à l'écoute des Français de l'étranger et qui sait comprendre leurs attentes et leurs spécificités.

en plus du vote à l'urne et du vote électronique, le recours au vote par correspondance sous pli fermé pour les prochaines élections consulaires.

Il était donc très important de reprendre cette possibilité de vote par correspondance dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. En effet, nous n'avons aucune idée de ce que sera la situation sanitaire en mai 2021 dans certains pays. Il faut songer que le vote électronique n'est pas encore entré dans les moeurs de tous et suscite encore parfois de la méfiance chez certains de nos compatriotes. Or se rendre à l'urne, surtout lorsqu'il faut parcourir plusieurs heures de route, route, voire prendre un avion pour aller voter, ce qui arrive souvent pour les Français de l'étranger, peut, dans un contexte sanitaire dangereux, s'avérer impossible ou, à tout le moins, dissuasif.

La crise sanitaire qui touche tous les continents a démontré le rôle de ces élus, qui ont apporté un soutien absolument essentiel aux postes diplomatiques sous tension pour organiser les nombreux retours en France.

Cet amendement tend à autoriser, si la situation sanitaire dans le monde le permet, bien entendu, et sous réserve de l'avis du comité scientifique, la tenue des élections consulaires plus plus tôt- de préférence, au plus vite -, pour éviter un retard considérable de l'exercice de la démocratie locale. Quel

prochain, mais nous ne le saurions pas davantage en décembre ou en septembre ... Au fond, nous cherchons à nous donner un temps raisonnable pour permettre l'organisation du scrutin, quelle que soit la situation sanitaire.

nous souhaitons que le vote par correspondance puisse être organisé dans des conditions de sécurité qui évitent toute fraude. En tout état de cause, notre devoir est de choisir la date des élections consulaires. Nous ne pouvons pas laisser au Gouvernement le soin de choisir cette date, au moment

aux Français qui vivent hors de France et à tous ceux qui vont se présenter la sécurité et la stabilité qui permettent une campagne électorale sereine. Bien entendu, on peut toujours envisager le pire, c'est-à-dire que la catastrophe que nous avons vécue ces derniers mois se reproduira l'année prochaine,

Cet amendement prévoit que le Gouvernement remette à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE), au plus tard trois mois après la promulgation du texte, c'est-à-dire juste avant la réunion de l'AFE qui aura lieu au mois d'octobre, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.

des conseillers des Français de l'étranger, ce qui permettrait d'habituer nos compatriotes établis à l'étranger à cette nouvelle dénomination. Par ailleurs, les dispositions de cet amendement prévoient que la fonction

que les conseils consulaires soient présidés par un élu, et c'est heureux, à compter du prochain renouvellement général des conseillers consulaires qui devait avoir lieu en mai 2020. 2020. Le présent projet de loi prévoyant le report des élections consulaires à mai 2021, la commission des lois du Sénat a fort heureusement proposé, à l'article 4, de 4, de ne pas attendre 2021 pour l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi n° 2019-1461. La date du 1 octobre 2020 retenue visait à laisser à nos postes consulaires le temps de s'organiser. Certains conseils consulaires risquant cependant de procéder à l'élection de leur président dès septembre, il semble opportun de ne pas attendre le 1 octobre et de prévoir une entrée en vigueur dès la promulgation

le rôle des conseils consulaires dans l'application du plan d'urgence pour les Français de l'étranger. Doivent-ils se prononcer sur les aides sociales ?

... Les conseillers consulaires sont des élus locaux et des Français de l'étranger. Ils perçoivent à ce titre une indemnité, qui est calculée sur la base de l'indemnité mensuelle de référence d'un conseiller municipal d'une circonscription d'environ 100 000 habitants, habitants, majorée au titre de l'expatriation, et à laquelle s'applique un indice de base permettant de tenir compte des disparités du coût de la vie dans les différents pays. Ce calcul ne prend cependant aucunement en compte la dimension de la circonscription que les conseillers consulaires ont à couvrir- parfois plusieurs pays -ni la taille de la communauté française qu'ils ont à représenter, ce qui crée des inégalités entre les élus et nuit souvent au bon exercice de leur mandat. Cet amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement sur ce sujet avant la tenue des prochaines élections des conseillers consulaires de l'étranger. Quel

peut être éligible au remboursement de ses frais sur une base forfaitaire si le coût de ses déplacements de l'année représente plus de 60 % du montant annuel de son indemnité. Si je comprends l'intention de Mme la sénatrice, un certain nombre de dispositions existent d'ores et déjà.

on en a parlé dès le début de nos travaux -, à l'approche du second tour, l'évolution de la situation sanitaire dans certaines communes, comme l'apparition de, ne permette pas le maintien de l'élection dans lesdites communes. Il tend à réintroduire la convocation du nouveau scrutin par arrêté du préfet de département compétent en lieu et place d'un décret en conseil des ministres. Je ne vous cache pas que j'ai été surpris de voir que votre assemblée, qui représente pourtant les collectivités locales et défend

Au-delà de cette question de forme, l'amendement vise à rétablir la prorogation du mandat des conseillers municipaux dans les communes qui seraient concernées par l'annulation du second tour jusqu'au terme du nouveau scrutin, et non jusqu'au 31 octobre. En conséquence, la première réunion de l'organe délibérant des EPCI mixtes se tiendrait au plus tard le quatrième vendredi suivant le premier tour du nouveau scrutin, et non le 20 novembre.

Ce n'était pas l'objet de l'argumentaire présenté par le ministre, mais c'est la motivation principale de la modification que nous avons apportée

de prévenir son ministre de la convocation des électeurs et que, au fond, à partir du moment où le ministère serait impliqué dans la décision du préfet, ce ne serait pas beaucoup plus compliqué de s'en tenir au droit commun, c'est-à-dire la

Projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. » Voici quel sera

Merci,